La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 29 septembre 2016 a été publié sur le site

du décès de notre ancien collègue Michel Rigou, qui fut sénateur de la Charente-Maritime de 1980 à 1989. J'ai également appris il y a quelques jours, comme vous tous, le décès de notre ancienne collègue Marie-Thérèse Goutmann, qui fut sénatrice de Institutrice puis directrice d'école, Marie-Thérèse Goutmann s'engage dans les rangs du parti communiste français, militant notamment pour des causes qui lui tenaient à coeur, telles que celles des femmes, des droits de l'enfant ou encore de la paix en Algérie.

devenant ainsi la première femme à présider un groupe parlementaire. Au sein de notre assemblée, elle poursuit ses combats pour les femmes : elle dépose de nombreuses propositions de loi visant, par exemple, à financer la construction de crèches ou à protéger les femmes enceintes contre les licenciements abusifs.

En application de l'article 5 de notre règlement, j'ai reçu les déclarations des présidents des groupes qui souhaitent être reconnus comme groupes d'opposition ou groupes minoritaires au sens de l'article 51-1 51-1 de la Constitution. M. Didier Guillaume, président du groupe socialiste et républicain, a fait connaître que son groupe se déclare comme groupe d'opposition. M. François Zocchetto, président du groupe UDI-UC, Mme Éliane Assassi, présidente du groupe communiste républicain et citoyen, M. Jacques Mézard, président du groupe du RDSE, et M. Jean Desessard, président du groupe écologiste, ont quant à eux fait savoir que leurs groupes se déclarent comme groupes minoritaires. Chacun de ces groupes pourra donc, au cours de la session, bénéficier des droits attribués aux groupes d'opposition et minoritaires par la Constitution et notre règlement, notamment dans le cadre des « espaces » qui leur sont réservés. En application de l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l'examen du projet de loi ratifiant les ordonnances du 14 mars 2016 relatives à la partie législative du code de la consommation et du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'égalité et à la citoyenneté

Monsieur le président, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs,

Des forces centrifuges sont à l'oeuvre, la fragmentation nous guette collectivement. Des années de crise économique, l'épreuve sans précédent du terrorisme fragilisent notre capacité à vivre en commun. La République n'est pas une République n'est pas une statue de cire. Elle est vivante ; elle s'adapte ; elle évolue. À chaque époque, elle doit se reformuler. Nous vivons une époque où ce que nous pensions inébranlable ne l'est peut-être pas tant que cela

faire bloc quand rodent les semeurs de désordre et les prédicateurs de lendemains qui pleurent. Il n'y a pas de prophétie plus auto-réalisatrice que celle qui stipule que le progrès a pris fin,

J'irai à l'essentiel. La citoyenneté, c'est ce qui caractérise l'appartenance à la communauté nationale ; ce sont des droits, essentiels, et des exigences. Notre pays est riche des engagements de ses citoyens : 23 millions de Français adhèrent à une association ; 16 millions sont des bénévoles actifs, l'engagement des trois quarts d'entre eux ayant un

de ce que j'ai pour habitude d'appeler la « culture de l'engagement », nous allons créer la réserve civique, pour que chacun puisse occasionnellement se mettre au service de l'intérêt général. Les événements tragiques de 2015 et de 2016 ont montré que nos concitoyens cherchent à aider dans des moments de crise, sans trop savoir comment faire. Ils pourront désormais devenir réservistes civiques, mobilisables pour aider des personnes sinistrées à la suite d'inondations, en appui de ceux qui accompagnent les personnes âgées en cas de canicule, pour nettoyer des plages après une pollution ou pour faire vivre les valeurs de la République sur un territoire en difficulté. Le projet de loi, tel qu'il était issu des travaux de l'Assemblée travaux de l'Assemblée nationale, créait un congé d'engagement non rémunéré de six jours fractionnables. La commission spéciale du Sénat a décidé de supprimer cette disposition ; j'en prends acte et je le regrette. Nul ne peut nier ici que ce gouvernement est attentif aux entreprises de ce pays. Elles sont essentielles à la reprise, mais l'engagement citoyen ou associatif l'est tout autant. Les actifs rencontrent des difficultés pour s'engager ; le congé d'engagement y répond, pour que le bénévolat actif ne soit pas réservé à ceux qui ne travaillent pas.

C'est la raison pour laquelle nous allons donner un nouvel élan au service civique, outil du lien social. C'est d'ailleurs une proposition de loi déposée au Sénat en 2009 par Yvon Collin qui est à l'origine de la loi de 2010 relative au service civique. Vous le savez, le Président de la République a fixé un objectif ambitieux.

Nous consolidons également des dispositifs facilitant l'accès des jeunes à leur autonomie. Ainsi, en matière de santé, nous renforçons le droit à une information complète sur les droits relatifs à la couverture maladie. Nous vous proposerons en outre, dans ce cadre, de rétablir la sécurisation du dispositif de la CMU-C pour les jeunes en rupture familiale ; cette mesure a toute sa place dans ce texte. L'autonomie, c'est aussi la mobilité. Beaucoup d'entre vous représentent ici des territoires ruraux. Vous savez combien, sans permis de conduire, tout devient difficile. Je veux saluer ici les avancées obtenues à cet égard. Il sera désormais possible, grâce à ce projet de loi, de mobiliser le compte personnel formation pour financer la formation au permis de conduire.

Je regrette que la commission spéciale du Sénat ait supprimé la possibilité, pour les mineurs de 16 ans et plus, de devenir directeur de publication, la prémajorité associative ou le droit de demander son émancipation à 16 ans. la loi de 1901 n'a posé aucune condition d'âge pour créer une association, sans que cela soulève de difficultés en matière de responsabilité des mineurs. Je n'oublie pas que c'est le Sénat qui, en saisissant le Conseil constitutionnel en 1971, sauva la liberté d'association telle que nous la concevons aujourd'hui.

leur permettre d'aller progressivement vers leur majorité. C'est l'apprentissage de la responsabilité, l'apprivoisement de la citoyenneté. J'invite donc le Sénat à faire sienne la phrase de Fénelon

Elles ont pourtant une cohérence, en ce qu'elles participent à faire vivre la promesse de l'égalité républicaine partout et pour tous. En tant que ministre de la ville, je suis surpris que les dispositions sur le droit d'interpellation des conseils citoyens aient été supprimées par la commission spéciale.

Nous renforçons également notre arsenal de lutte contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme et tout ce qui, subrepticement ou bruyamment, altère chaque jour un peu plus le lien social. Nous généralisons la circonstance aggravante de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie et de sexisme. Le projet de loi tend aussi à améliorer la répression des délits de provocation et d'injures racistes ou discriminatoires, en renforçant les peines encourues, en ajoutant la peine de stage de citoyenneté et en levant les obstacles juridiques

de faits qui mériteraient condamnation. Si, en la matière plus qu'en tout autre, nous avons un devoir moral d'efficacité, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est de celles que l'on touche avec une main prudente. La commission spéciale a adopté plusieurs amendements qui bouleversent les grands équilibres de cette loi protectrice de la liberté d'expression. Pour sa part, le Gouvernement est attaché aux garanties procédurales prévues par la loi de 1881 ; je ne doute pas que nos débats seront riches sur ce point. Je pourrais évoquer encore de nombreuses autres dispositions. Le texte a été, selon l'expression consacrée, considérablement enrichi au cours de son examen à l'Assemblée nationale.

Je connais la tempérance du Sénat, son souci de la précision, sa rigueur, son exigence. Je sais aussi que cette tempérance peut être audacieuse,

à mon tour je souhaite vous présenter l'une des briques du grand édifice du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté. L'ambition de ce texte est grande, car il s'agit d'une mobilisation générale pour le vivre ensemble, ce ciment indispensable de notre pacte républicain. À l'heure où la tentation du repli sur soi s'accroît, où la peur de l'autre grandit, nous devons tout faire pour redonner confiance à nos concitoyens. Nous avons l'immense responsabilité de ne pas nous laisser envahir par ce mouvement insidieux de défiance de tous et de trouver des réponses pour favoriser la cohésion sociale dans notre pays. J'en suis convaincue, la manière dont nous faisons société se traduit avant tout dans la manière dont nous partageons l'espace public dans toutes les villes, tous les quartiers et tous les territoires. Depuis la loi Siegfried de 1894, le modèle français du logement social s'est imposé comme un pilier de notre pacte républicain, au même titre que la sécurité sociale et les services publics. Ce modèle généraliste, qui permet de réconcilier droit au logement et mixité sociale, doit être sans cesse renforcé et amélioré, car il est une force inouïe pour notre pays, regardé par nombre d'autres pays européens. Je le redis, le logement social est le logement de tous, 70 % des Français y étant éligibles. Pendant longtemps, et en particulier après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a fallu construire vite et beaucoup, nous nous sommes contentés de cet impératif d'efficacité.

: ce qui devait être un urbanisme de rêve, sans voitures, avec un espace pour chaque fonction, s'est mué en lieu de relégation sociale. La diversité sociale, clef du succès de ces quartiers, s'est peu à peu estompée. Oui, nous avons construit vite, trop vite parfois, souvent de manière trop indifférenciée, pour répondre à l'urgence. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce que le Premier ministre a appelé, après les attentats de janvier 2015, l'« apartheid social et territorial Ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité dans de nombreux quartiers. Cette situation est la résultante de logiques d'exclusion par le haut et par le bas. Certains entretiennent en effet sciemment une ségrégation spatiale, par le refus délibéré de prendre leur part dans la solidarité nationale, notamment en ne construisant pas de logements sociaux : s'il y a des ghettos de pauvres, c'est aussi parce qu'il y a des ghettos de riches. C'est la résultante de logiques urbaines ayant conduit à construire des logements, mais pas les équipements publics et les transports en commun qui permettraient de relier certains quartiers ouverts au reste de l'agglomération. C'est la résultante, enfin, de logiques discriminatoires -n'ayons pas peur des mots -qui enferment des jeunes de talent dans leur quartier, parce qu'on leur refuse ici un entretien d'embauche, là l'accès à un logement au-dehors de leur quartier, au motif que leur nom de famille a une consonance qui ne plaît pas. Nous avons toutes et tous une responsabilité dans cet empilement de difficultés qui entretiennent le repli sur soi et la défiance. Nous avons surtout le devoir d'y remédier, car, ne nous y trompons pas, le fléau de la discrimination n'affecte pas que ceux qui en sont victimes : c'est la société tout entière qu'il fissure en profondeur. Il nous faut pour ce faire reprendre le flambeau d'une politique du logement qui, historiquement, a constitué un moteur essentiel et reconnu de tous du progrès social dans notre pays.

Récemment, l'État a tenu ses engagements et sécurisé le financement du logement social, avec les prêts de haut de bilan, accordés aujourd'hui à l'ensemble des bailleurs sociaux, la création du Fonds national des aides à la pierre et la réforme d'Action logement, que j'étais venue défendre devant vous.

sociale. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous n'avez ni repris ni amélioré cet équilibre entre droit au logement et mixité sociale, entre objectifs d'intérêt général et nécessaire adaptation aux situations locales.

En supprimant la possibilité automatique, pour les préfets, de procéder à des attributions si les collectivités, les bailleurs ou les réservataires ne respectaient leurs objectifs de mixité sociale, vous avez limité la nécessaire pression nationale et la capacité d'intervention de l'État qui en est l'indispensable moteur. Enfin, en supprimant l'obligation, pour les bailleurs, de publier la liste de leurs logements vacants, vous avez réduit un objectif de transparence visant à faire des demandeurs de logement social les acteurs de leur recherche de logement.

Au travers du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, le Gouvernement a souhaité consolider les fondements de son périmètre d'application, pour le rendre plus cohérent avec la réalité du terrain et renforcer les moyens opposables aux communes qui s'exonèrent de l'effort national de solidarité. Peut-on réellement vouloir agir à rebours de ce mouvement, alors que, aujourd'hui, on peut vivre en France dans une agglomération urbaine tout en étant coupé du monde, alors qu'on peut vivre dans des quartiers totalement relégués ?

Je le redis ici, ce qui fonde ce projet de loi, c'est le renforcement des « ressorts » du vivre ensemble, grâce à des logiques de solidarité qui doivent s'imposer à toutes et tous, car elles profiteront, en fin de compte, à toutes et à tous.

Pourtant, je connais votre implication dans vos territoires. Certaines et certains d'entre vous se battent pour des villes plus inclusives, au service de celles et de ceux qui vivent parfois hors des circuits de la vie sociale.

C'était le sens de l'article 20 du projet de loi, qui prévoyait une réforme ambitieuse des attributions de logements sociaux. Ainsi, nous souhaitons que 25 % des attributions de logements sociaux à l'échelle de l'intercommunalité soient réalisées au bénéfice des 25 % de demandeurs les plus modestes.

Le texte que la commission spéciale du Sénat a adopté revient sur l'ensemble de ces dispositions : moins de transparence, moins d'obligations pour les collectivités en termes de mixité sociale ou de production de logements sociaux. Je le dis solennellement devant vous, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs : on ne peut dresser la mixité comme le paravent de l'exclusion. Refuser un logement à un ménage prioritaire dans un quartier de la politique de la ville revient à le laisser sans solution. C'est surtout renoncer au respect élémentaire du droit au logement. Telle n'est pas ma vision ! Je veux au contraire ouvrir tous les quartiers à tous les ménages. Le gouvernement auquel j'appartiens entend faire prévaloir dans le logement social un droit positif et un droit d'accès, et non un droit de séparation ou d'exclusion. Telle est la substance première de ce titre II relatif à la mixité sociale dans le logement. Le Gouvernement défend en outre, au nom de l'efficacité des politiques publiques, un pacte territorial renforcé entre État, collectivités, bailleurs et usagers. Il vise aussi à promouvoir une République en actes. N'oublions jamais que l'autonomie, la réussite scolaire ou encore l'accès à un emploi sont intimement liés à l'accès à un logement digne. Avoir un chez-soi, au-delà d'un simple toit, c'est une exigence quotidienne pour des millions de nos concitoyens ; y répondre requiert notre mobilisation J'aurais aimé que nous puissions être unis au service de cette nécessité. Je constate que ce n'est pas le cas. J'en prends acte, mais je serai présente pour défendre, mesure après mesure, amendement après amendement, des dispositions que je crois essentielles à l'affirmation du pacte républicain.

et de la question terrifiante qu'ils ont posée à toute la Nation- comment des enfants de France peuvent-ils avoir pour seul dessein sa destruction ? -, le projet de loi « Égalité et citoyenneté » répond à l'objectif ambitieux de renforcer la cohésion de la société française en encourageant l'engagement civique- tout particulièrement celui des jeunes, en les accompagnant vers l'autonomie -et en luttant contre les discriminations. Les titres I et III de ce texte, que je suis chargée de rapporter, pourraient rassembler, autour de ce constat alarmant d'une désintégration de notre société, laquelle n'a cessé d'ériger en valeurs suprêmes la liberté et les droits individuels, au détriment de la responsabilité et de la solidarité réelle.

destinées à renforcer l'appartenance républicaine, affirmant avec raison que la nation française constitue un héritage à partager, qu'il nous appartient de faire vivre et de transmettre.

législatif, en quelque sorte traitant de sujets aussi divers que les cantines, les ordonnances de Charles X ou les auberges de jeunesse. II a tant dérivé que, dans l'exercice de ma mission de rapporteur, j'ai eu à plusieurs reprises l'impression de perdre le fil du propos initial, tout comme, d'ailleurs, j'ai perdu de vue, au cours de l'été, la secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle

Ainsi, le service civique universel est une chimère, sachant que l'État peinera déjà à accueillir en service civique la moitié d'une classe d'âge à la fin de 2017 et au début de 2018. Troisièmement, nous devions supprimer les dispositions relevant du pouvoir réglementaire et les très nombreuses demandes de rapport.

devions affirmer notre rôle de législateur responsable en refusant que le Sénat soit une simple chambre d'enregistrement. C'est le sens de notre proposition exigeante de contrôle renforcé et sécurisé de la procédure d'ouverture d'une école.

à mettre fin à ce qu'il appelle « l'emballement législatif et réglementaire », qui produit chaque année un million de mots supplémentaires. Fidèles à cette ligne de conduite,

Permettez-moi d'exprimer, avec beaucoup de respect, un réel étonnement. Si des délits d'entrave numérique à l'IVG sont effectivement constatés et d'ampleur,

Sous-entendre que la décision de la commission spéciale constituerait la trahison d'une femme d'exception, Simone Veil, est indécent, détestable et indigne. Simone Veil, ministre centriste, a suscité l'engagement en politique de beaucoup de femmes. Je suis l'une de ces femmes, et je ne peux taire ma profonde indignation devant cette manoeuvre grossière de dénigrement, qui masque en réalité, mes chers collègues, une impréparation fiévreuse du Gouvernement et une tentative sans scrupule de rassembler une majorité quelque peu effritée ! Les Français

j'ai approuvé le souhait de mettre en oeuvre la refondation d'une société responsable et solidaire, car un pays n'a pas d'avenir sans l'engagement de tous ses citoyens. En ce sens, la réserve civique, le service civique, l'accès facilité à la fonction publique sont de justes dispositions. Mais je le redis, très calmement : ce texte a largement dérivé, tant et si bien que son esprit initial s'est évaporé. Notre estimable assemblée manquerait à son devoir si elle ne demeurait pas le lieu de la réflexion et du travail serein. Pour conclure, je veux remercier, pour leur active participation et leur esprit constructif, nos collègues de la commission spéciale, et saluer l'appui

Construire davantage de logements sociaux, loger mieux et en plus grand nombre les ménages modestes, défavorisés ou précaires, favoriser la mixité sociale et éviter la création de ghettos sont autant d'objectifs auxquels la commission spéciale et le Sénat tout entier s'associent, et ce depuis longtemps. Très bien ! Cependant, si nous partageons ces objectifs, nous ne partageons pas la méthode choisie par le Gouvernement.

Les différences considérables existant entre les départements, d'ailleurs plus marquées encore à des échelles plus fines, montrent que les problèmes du logement ne doivent pas être traités globalement, mais au cas par cas, au cas par cas, au rebours des lois conçues et votées depuis Paris. La confiance dans les élus locaux et le réalisme des dispositifs proposés ont guidé la commission spéciale dans ses choix sur ce volet. Tout d'abord, le projet de loi prévoit de renforcer la mixité sociale dans le logement en diversifiant de façon plus volontariste les attributions de logements, de manière que les ménages les plus modestes ne soient pas systématiquement orientés vers les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Autre problème, cette politique risque fort d'être ingérable. En effet, vouloir influer sur les politiques d'attribution pourrait conduire à des condamnations pour discrimination.

la vie que des liens sociaux qui les unissent à leurs anciens quartiers et qui représentent autant de ressources négligées par les approches techniciennes. C'est pourquoi la commission spéciale a proposé que ces objectifs soient déterminés par accord entre les collectivités locales concernées et le préfet. Mettre en place des objectifs déconnectés de la réalité et sanctionner leur non-réalisation par une substitution automatique du préfet à la collectivité comme le propose le Gouvernement, ne peut que décourager les maires de construire des logements sociaux ou d'apporter leur garantie aux organismes qui les construisent. Tout à fait les délégations du contingent préfectoral, la possibilité de créer une commission d'attribution ou la voix prépondérante du maire sont autant d'éléments qui incitent les maires à maintenir leurs engagements en matière de logement. Pour tenter d'augmenter l'offre locative sociale, le projet de loi prévoit de renforcer les contraintes imposées par la loi SRU. La dimension productiviste a progressivement pris le pas sur le volet qualitatif de la loi SRU, renforcé par la loi ALUR, laquelle a resserré l'étau autour des communes contrevenantes. Or chacun sait que les obligations inscrites dans la loi sont intenables. Le Gouvernement n'a pas voulu revoir les modalités d'application de cette loi et s'est contenté d'introduire deux nouvelles exemptions et de renforcer les pénalités financières à l'encontre des communes déficitaires ou carencées. Au contraire, la commission spéciale a souhaité redéfinir l'ensemble du dispositif de la loi SRU, non pas, comme j'ai pu l'entendre dire, pour exonérer les communes de leurs obligations de construction de logements sociaux, mais simplement pour permettre une meilleure adaptation de l'objectif aux réalités du terrain, dans un souci d'efficacité et de bonne gestion, et pour éviter un effet d'éviction trop important de l'offre privée. Ainsi, un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le maire et le préfet permettra de déterminer, en fonction de la situation locale, le taux de logements sociaux et surtout l'échéance à laquelle ce seuil devra être atteint. De même, dans un contexte de baisse des dotations, la commission spéciale a considéré

Considérant qu'il ne fallait pas ignorer la question de la mixité sociale dans les communes ayant plus de 50 % de logements sociaux, la commission spéciale a proposé la mise en place d'un contrat d'objectifs et de moyens leur permettra de diversifier leur offre de logements par la construction de logements intermédiaires. S'agissant, enfin, des gens du voyage, la commission spéciale a cherché à répondre aux difficultés rencontrées par les élus locaux. Sans remettre en cause les droits nouveaux accordés aux gens du voyage, elle a simplifié et modernisé les procédures d'évacuation des campements illicites situés dans les communes remplissant leurs obligations d'accueil. Très bien ! La commission spéciale vous propose, mes chers collègues, d'adopter ce texte, au bénéfice des modifications apportées.

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, que peut-on attendre d'un gouvernement dont l'une des ministres estime que « la société française est d'abord minée par le repli identitaire » Comme plusieurs millions de Français, je crois au contraire que la société française est d'abord minée par le fait que notre pays et notre société sont infiltrés par des ennemis de la France ! Que proposez-vous ? Votre politique peut se résumer ainsi : « Le vivre-ensemble décrété est un échec ; décrétons-le » Pour faire avancer votre idéologie et faire taire ceux qui pensent différemment, vous n'hésitez pas à flirter avec le totalitarisme, si j'en crois, par exemple, votre amendement n° 664, vos mesures pro-migrants imposées à nos concitoyens, ou encore votre souhait de retirer aux maires des prérogatives en termes de logement. Certes, période préélectorale oblige, la majorité sénatoriale est revenue sur les mesures les plus idéologiques, mais c'est bien l'ensemble des politiques menées depuis des décennies qui ont abouti à la situation que nous connaissons aujourd'hui, prophétisée par les patriotes que la classe politique a préféré vilipender pendant des années. Ainsi, au nom du vivre-ensemble, vous avez créé le communautarisme ; au nom de la lutte contre le racisme, vous avez créé des individus qui rejettent la France, ses valeurs, son histoire ; au nom de la mixité sociale, vous avez créé des ghettos.

Il passe par une réflexion sur notre identité, sur nos racines et sur notre futur. Il passe par la volonté de transmettre l'amour de la France et de sa civilisation bimillénaire, par la volonté de préserver nos spécificités alors que le risque de l'uniformité guette notre planète, et, bien sûr, par le retour à une pleine et entière souveraineté du peuple français. de parler de citoyenneté, il faut remonter à la notion qui lui est liée : la nationalité ! Une profonde remise en cause du code de la nationalité me semble un préambule nécessaire pour parvenir à lutter contre « l'apartheid territorial, social et ethnique », pour reprendre les mots du Premier ministre. De la nationalité découle la citoyenneté, avec ses droits et ses devoirs. Pour ce qui est des devoirs, cela commence par le respect des symboles de notre pays, en particulier son drapeau et son hymne. Nous présenterons ainsi un amendement visant à doubler les peines sanctionnant ceux qui outragent ces attributs de la nation. Pour ce qui est des droits, je propose leur renforcement ! Oui, il faut renforcer les droits des citoyens français, et le premier de ces droits, c'est que les Français soient, en France, servis en priorité ! C'est scandaleux ! La priorité nationale, dans tous les domaines- logement, emploi, aides sociales, etc. -, est le premier des droits qu'il faut renforcer pour reprendre des mots contenus dans ce texte, « encourager l'engagement républicain de tous les citoyens pour faire vivre la fraternité » ! La première idée à développer, pour faire vivre le sentiment d'appartenance à la nation française, est que le pays doit s'occuper en priorité, ce qui ne veut pas dire en exclusivité, des fils et des filles de France France ? L'existence même de ce projet de loi est un aveu de l'échec de vos politiques. Je vous en prie, n'essayez pas de réparer vos erreurs, d'autant que vous n'êtes pas prêts à remettre en cause l'idéologie qui a précisément eu pour conséquence la situation que nous connaissons. Laissez la place à ceux qui veulent servir les Français, à ceux qui veulent faire vivre la nation française, à ceux qui veulent que la civilisation française continue de briller dans le monde, bref à ceux pour qui, selon les mots d'un lieutenant tombé au champ d'honneur, « France n'est pas un vain mot

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, près de dix-huit mois après l'attentat contre, le projet de loi « Égalité et citoyenneté », qui avait été annoncé comme une réponse de l'État aux fractures de notre société, nous est présenté. Je dois dire la difficulté d'appréhender ce texte, tant il lui manque l'essentiel, c'est-à-dire un fil directeur et une ambition, une structure et une cohérence. Ce projet de loi se présente comme une accumulation de mesures, dont la portée et la pertinence sont aléatoires, voire contradictoires. Cela entache sa lecture et sa compréhension.

tout comme il n'y a pas de citoyenneté sans égalité, puisqu'au coeur de la notion de citoyenneté se trouve celle d'égalité de tous les citoyens, porteurs des mêmes droits et des mêmes devoirs.

La citoyenneté, c'est ce qui fait bien commun entre les individus ; c'est ce que l'on appelle, en droit, « l'intérêt général ». Cette notion fonde l'existence des services publics et de la fonction publique pour garantir le respect des droits acquis pour tous, ciment de la République. Or il n'est pas question de cela dans ce texte. Pis, ce qui est désigné comme la source des maux de notre société, ce n'est pas la pauvreté et l'exclusion, les écarts de richesse et la reproduction des inégalités : c'est la concentration de cette pauvreté dans quelques quartiers. L'objectif défini n'est donc pas de s'attaquer à la pauvreté, mais de mieux la distiller sur le territoire, de la rendre moins visible, et donc plus acceptable. Pour ce faire, le Gouvernement recourt aux notions aléatoires d'« égalité des chances » et de « mixité sociale l'exécutif, sans surprise, s'inscrit donc dans une logique de gestion de la pénurie plutôt que dans une volonté réellement transformatrice. Étonnamment, ce projet de loi n'aborde la question de l'« entre soi » qu'au travers du prisme du logement social et des quartiers populaires, comme si l'« entre soi » n'existait pas dans d'autres quartiers, comme si seules les couches populaires étaient concernées par la perte de sens et de valeurs. C'est oublier un peu vite d'autres formes de comportements antirépublicains, comme la fraude fiscale, la corruption, la délinquance en col blanc.

S'appuyant sur ces ambiguïtés et ces lacunes, la commission spéciale a totalement récrit ce projet de loi, en y apportant de la cohérence. Malheureusement, cette cohérence est avant tout celle du rejet de toute contrainte, de toute règle, sous couvert de défense de la libre administration des collectivités et de la liberté des entreprises,

Nous avons ainsi assisté à un « détricotage » total du droit au logement. La loi SRU a été vidée de sa substance, alors même que le nombre de demandeurs de logement ne cesse d'augmenter et que le mal-logement progresse. Pis, les nouvelles dispositions pénalisent même les maires bâtisseurs, en les obligeant à construire du logement privé plutôt que du logement public. Les valeurs portées par la majorité sénatoriale de droite ont envahi ce texte, une société du chacun pour soi, une société où les droits sont à la carte, changeant au gré du lieu de résidence, une société qui favorise l'« entre soi » et la reproduction des inégalités. Les élus communistes et républicains, pour leur part, portent un tout autre diagnostic et ont une tout autre ambition pour notre pays. Le problème des quartiers populaires, c'est non pas leurs habitants, mais bien les politiques nationales qui y ont été menées. Le problème, c'est l'effacement de l'État par la suppression des services publics, le manque de fonctionnaires, le niveau record du chômage des jeunes, le recul de l'école comme catalyseur de l'égalité, tout cela engendrant un sentiment dangereux d'abandon. Nous vivons dans une société de plus en plus inégalitaire, une société marquée par les reculs sociaux, où l'on veut nous faire croire que la précarité serait une fatalité, une société où l'ascenseur social est bloqué, où le déclin est présenté comme inexorable.

esprit, les dénis de démocratie, le recours répété au 49.3, le non-respect de la parole politique ont fini de miner l'idée d'une République du peuple au service du peuple. L'interférence des intérêts privés avec les politiques publiques la faiblesse des modèles de représentation ont ruiné l'idée même que la politique pouvait être la source d'un progrès collectif, et non simplement l'outil de reproduction d'une élite autoproclamée. une identification erronée des problèmes et des maux de notre société, ce projet de loi ne peut y apporter les bonnes réponses. Le retour de l'État et la « République en actes » promis par le Premier ministre, être aussi le retour des services publics, leur modernisation, leur diversification, pour mieux répondre aux besoins d'une société moderne ouverte sur le monde, d'une société humaine. Ainsi, nous estimons que la responsabilité première des pouvoirs publics devrait être de redéfinir ce qui nous rassemble

En étant focalisé sur les jeunes et les quartiers, ce texte, tel que récrit par la droite, participe au brouillage idéologique, aux amalgames et à la stigmatisation. Voilà, mes chers collègues, l'état d'esprit dans lequel nous abordons cette discussion : nous avons le sentiment, une nouvelle fois, d'une occasion manquée, alors même qu'il y a urgence à édifier une société apaisée,

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, tortueux et long est le chemin qui doit mener de l'égalité formelle, proclamée dès 1789, à l'égalité réelle, tant promise mais si difficile à atteindre.

La recherche de l'égalité des droits et la valorisation de la citoyenneté doivent sous-tendre toute politique gouvernementale, et il est encourageant que ces deux objectifs Si l'on peut regretter que ce texte revienne sur des lois récemment adoptées ou rejetées par le Parlement, je tiens à saluer le travail de nos deux rapporteurs. Il a permis de recentrer quelque peu le texte et de lui redonner une cohérence qu'il n'avait pas ou plus.

du taux de ménages les plus démunis à loger en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il ne faut pas exonérer d'une telle obligation les collectivités ayant la capacité de la remplir.

Mes chers collègues, il n'est pas aisé de trouver l'équilibre idéal entre l'objectif de l'égal accès de tous au logement et celui de mixité sociale. Des efforts restent à accomplir ; nous y reviendrons. la politique en faveur de la jeunesse, notre groupe se réjouit, en particulier, de la montée en puissance du service civique. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, c'est une proposition de loi du RDSE, déposée sur l'initiative d'Yvon Collin, qui a donné naissance au service civique. Le projet de loi que vous nous présentez en poursuit la construction, développant la diversification des structures d'accueil, étendant l'accès du dispositif aux étrangers et prévoyant la reconnaissance de cet engagement dans l'enseignement supérieur ou au titre des concours de la fonction publique. Si certaines dispositions visent à accompagner les jeunes dans l'exercice de leur citoyenneté ou à encourager leur participation plus active à la vie de la cité, elles cachent parfois l'incapacité des gouvernements successifs à garantir à une jeunesse de plus en plus précarisée des conditions d'existence dignes : un toit, une éducation de qualité, un emploi. Malgré les efforts déployés, une partie des jeunes ne s'en sort pas.

Par ailleurs, je partage la volonté du Gouvernement de renforcer les contrôles sur l'instruction à domicile et les établissements privés hors contrat. Sans qu'il s'agisse pour nous d'entraver la liberté d'enseignement et la liberté pédagogique, je soutiendrai des amendements en ce sens. outre le contrôle sur l'instruction dispensée aux enfants, il convient de vérifier par un contrôle médical qu'il n'y a pas, par exemple, de signes d'isolement, de désocialisation, de mauvais traitements ou d'influence sectaire. Certes, les dérives ne sont pas majoritaires, mais elles existent et doivent être combattues avec force, dans l'intérêt de l'enfant et de la défense des valeurs de la République. Je regrette donc que nos amendements aient été frappés d'irrecevabilité financière alors que le gage a été levé sur d'autres amendements impliquant pourtant une augmentation indispensable des moyens de l'inspection

lutte contre les inégalités doit commencer sur les bancs de l'école. Depuis quinze ans, des études nous alertent sur la panne de l'ascenseur social à l'école. C'est le plus grand défi que nous devons relever, avec celui de l'emploi. Dans cette logique, nous devons rester vigilants. Les dispositifs proposés doivent profiter en priorité à l'école publique, plutôt qu'à l'enseignement privé, qui recueille les élèves les plus favorisés. Cette tendance nous éloigne totalement de l'objectif de mixité sociale. Mais, pour réussir, il faut d'abord convaincre. Comme l'exprimait très justement le très radical Édouard Herriot Une démocratie bien comprise n'est pas un régime qui maintienne artificiellement entre les hommes une égalité chimérique ; c'est un régime de libre sélection qui n'assigne d'autre limite à l'ascension sociale que les limites mêmes de l'effort et de la volonté de l'individu. Pour conclure, dans l'ensemble, ce texte contient des mesures positives, et d'autres plus incertaines. Mais, ce qui apparaît comme une évidence, c'est qu'il ne suffira pas à mettre un terme aux inégalités croissantes dans notre pays ; en la matière, la loi et la volonté politique ne peuvent suffire. C'est donc un travail de très long terme qui doit associer et engager l'ensemble des acteurs et, bien au-delà, des Français.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames les rapporteurs, ces deux dernières années ont été marquées par des événements particulièrement dramatiques, qui ont aussi montré l'ampleur des fractures sociales présentes dans notre pays et celle du sentiment d'abandon qu'éprouve une partie de la population. Exclusion sociale, marginalisation des personnes vulnérables, discrimination, non-accès aux droits : il est plus que temps de s'occuper prioritairement de remédier à ces fêlures profondes qui divisent et minent notre République. Le texte initial du Gouvernement contenait plusieurs propositions fortes. Malheureusement, de nombreuses dispositions phares ont été supprimées par la commission spéciale du Sénat, et le texte sur lequel nous travaillons aujourd'hui n'est pas du tout à la hauteur des enjeux.

qui a remplacé les objectifs chiffrés par une contractualisation au cas par cas. Les communes seront simplement tenues de ne pas passer sous la barre des 15 % de logements sociaux. Selon nous, c'est là une véritable régression, au regard de l'ampleur des besoins en matière de logement social.

de suivre de manière très opérationnelle le déploiement concret de ces mesures, des comités interministériels à la jeunesse, à l'égalité et à la citoyenneté ont été installés sous votre autorité, monsieur le ministre.

aux attentats du mois de janvier 2015 et à la réactivation, sous un jour nouveau, de fractures anciennes de notre société, le Gouvernement a fait de la réaffirmation et du rassemblement autour des valeurs de la République un objectif impérieux, au sein d'un plan d'ensemble que l'on peut intituler « La République en actes », concrétisé lors du premier comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté, au printemps de 2015. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, ce que souhaitent les jeunes aujourd'hui, c'est non pas seulement des mots, mais aussi des actes

Certaines de ces actions nécessitent une adaptation ou un prolongement législatif. Le présent texte est le complément nécessaire et pragmatique de l'action de l'État. de ce projet de loi, il s'agit donc d'aller plus loin dans la culture de l'engagement au service de l'intérêt général, de la société dans son ensemble et, prioritairement, de la jeunesse, en créant les conditions d'un parcours citoyen généralisé, depuis l'école primaire jusqu'à la terminale. La consécration en serait l'engagement dans le service civique, puis dans la réserve civique. Ce parcours sera matérialisé par un livret citoyen, remis à tous les jeunes dès l'âge de seize ans. Cet âge nous paraît d'ailleurs tardif pourquoi ne pas remettre le livret citoyen dès le cours préparatoire, afin que toutes les démarches citoyennes puissent effectivement y être consignées, à l'école, au collège, au lycée ? Le parcours citoyen généralisé soulève en outre la question de la valorisation de l'engagement dans le second degré. Pourquoi celui-ci serait-il réservé aux étudiants,

À ce sujet, nous ne pensons pas que les services de Bercy doivent garder le monopole de la définition du caractère d'intérêt général d'une association, même si cette reconnaissance a des conséquences fiscales. Il faut sortir la notion d'intérêt général de son sens strictement fiscal. Tout comme nous croyons à la pédagogie active- partir du faire pour maîtriser les concepts -, nous croyons à la citoyenneté active : s'impliquer dans un projet pour se sentir citoyen et développer des attitudes civiques. En parallèle des 300 heures d'enseignement moral et civique dispensées sur l'ensemble de la scolarité, développons au sein de l'école le débat démocratique, les projets citoyens, le tutorat par les pairs, pour plus de fraternité et de solidarité. Allons jusqu'au bout de cette démarche de promotion de la citoyenneté active en reconnaissant la prémajorité associative. Faisons confiance aux jeunes en leur permettant de construire de vrais projets associatifs en autonomie, en autogestion, oserai-je dire ! Le réseau national des juniors associations accompagne ainsi un millier d'associations de fait, créées et gérées par des mineurs. Oui, des mineurs sont présidents d'association, et cela ne crée pas de problème ! Oui, ils gèrent des budgets, sans difficulté majeure ! Alors, ne soyons ni frileux ni méfiants : le cadre formel d'une association est bien plus protecteur pour les mineurs que des pratiques informelles hors de tout cadre. Nous vous proposerons donc de rétablir l'article 15 , relatif à la prémajorité associative, et, dans le même esprit, l'article 15, sur l'extension du droit de publication des mineurs.

volet du titre II relatif à la mixité sociale dans l'habitat, les divergences au sein de notre assemblée sont également édifiantes. Le projet de loi était sous-tendu par l'ambition de mettre en place de nouveaux dispositifs pour assurer une meilleure répartition territoriale des attributions de logements En effet, les chiffres montrent une augmentation constante du nombre de ménages à faibles revenus dans les quartiers qui en comportent déjà une proportion importante. Réserver un quart des logements sociaux aux ménages les plus pauvres hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville a donc le mérite de mettre en oeuvre autrement la mixité sociale, avec des résultats rapidement évaluables. Le texte prévoyait également de poser les bases d'une réflexion intercommunale sur les attributions de logements sociaux, pour éviter les situations de blocage. Il donnait à l'État des moyens forts

Autre réponse apportée par le Gouvernement, toutes les communes nouvellement entrantes dans le dispositif de la loi SRU seront exonérées de prélèvements SRU pendant trois ans. En contrepartie de ces ajustements, le Gouvernement attend une contribution rigoureuse à l'effort de construction de logements sociaux sur les territoires où les besoins en logements sociaux existent. rebours de cette volonté, en commission spéciale, la majorité sénatoriale a vidé le dispositif de la loi SRU de son objet essentiel : la construction de logements locatifs sociaux sur tous les territoires. Mes chers collègues, est-ce vraiment le moment de réduire la pression en faveur de la construction de logements sociaux ? Pis encore, la commission spéciale a supprimé tout financement public pour la construction de nouveaux logements sociaux pour les communes qui en comptent déjà 50 % sur leur territoire. Cette mesure fait écho à celle qui a été prise au printemps par la région d'Île-de-France de mettre un terme au financement de logements très sociaux dans les communes qui en comptent déjà plus de 30 %. Mais, chers collègues de la majorité sénatoriale, que proposez-vous pour que les communes déficitaires se mettent enfin à construire des logements sociaux ?

Nous constatons d'ailleurs qu'une telle position ne fait pas l'unanimité dans vos rangs. Sans surprise, le groupe socialiste et républicain proposera de revenir à l'esprit du texte du Gouvernement sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Avant de conclure, je voudrais encore aborder deux points essentiels.

Actuellement, les actions de lutte contre l'illettrisme sont coordonnées avec succès par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, l'ANLCI. Parmi les mesures de la « République en actes » figure la création d'une agence de la langue française,

comme si elle voulait éviter de réitérer l'épisode de l'article 17 de la loi « santé », relatif à la suppression du délai de rétractation de sept jours en matière d'IVG. Nous savons tous que les femmes en détresse peuvent être manipulées par des groupuscules antiavortement,

Mes chers collègues, les mesures phare de ce projet de loi en matière de citoyenneté modèleront durablement notre société, si tant est qu'elles s'inscrivent dans une volonté politique durable. Durant le débat à venir, les sénatrices et les sénateurs socialistes n'auront de cesse de défendre les valeurs fortes portées par ce projet de loi, au nom de l'égalité et de la citoyenneté, solides piliers de notre République.

les attentats perpétrés sur notre sol depuis le mois de janvier 2015 ont effectivement été le révélateur des profondes fractures qui traversent aujourd'hui notre société. Les Français ont pris conscience qu'une partie de la jeunesse s'était peu à peu détachée de la République, vivant dans le déni de son appartenance à la communauté nationale et dans le rejet des valeurs qui fondent notre contrat social.

L'approche choisie par le Gouvernement sous-entend donc que les inégalités et le manque de mixité sociale sont en cause dans les phénomènes de radicalisation, de communautarisme et de rejet des valeurs républicaines. nous, le mal est, à l'évidence, bien plus profond. Les « territoires perdus de la République » souffrent aussi d'un laisser-aller de l'État, qui a trop longtemps accepté de voir son autorité bafouée et fermé les yeux sur les atteintes à l'ordre public et le repli communautaire. Quant à notre système scolaire, il ne remplit plus, depuis bien longtemps, son rôle de brassage, de transmission de notre langue, de notre culture et de notre récit national. Voilà pourquoi nous jugeons que la réponse proposée ici par le Gouvernement est bien trop parcellaire et passe à côté des véritables enjeux. Très bien ! Ce qui fait fondamentalement défaut à ce texte, c'est bien la réaffirmation d'un modèle envisagé dans sa globalité, c'est-à-dire avec ses droits et ses libertés, mais aussi avec ses devoirs et ses responsabilités, qui structurent le modèle républicain. Sans vision d'ensemble, ce projet de loi ne peut ni fixer de cap ni poser une réelle ambition. Deuxième défaut majeur de ce texte, il est devenu, au fil de la discussion, un véritable fourre-tout législatif, passant de 41 à 215 articles, égrenant des mesures disparates, oscillant souvent entre l'anecdotique et l'incantatoire, allant des questions d'alimentation durable aux règles de vente au déballage, du bizutage à la portabilité du lundi de Pentecôte, en passant par les gens du voyage et les langues régionales Ce matin même, en commission spéciale, nous avons examiné nombre d'amendements déposés dans la nuit par le Gouvernement et n'ayant, pour la plupart, aucun rapport avec l'objet du texte. Certains accusent le Parlement de lenteur : que l'on me permette de conseiller au Gouvernement de commencer par balayer devant sa porte Un texte censé répondre à un problème aussi grave que celui du délitement de notre pacte républicain ne peut pas être utilisé comme le dernier véhicule législatif avant le terminus de 2017. Fort heureusement, la commission spéciale du Sénat et ses rapporteurs se sont livrés à un important travail de toilettage, qui, à défaut de rendre ce texte décisif, le rend du moins plus acceptable en termes de procédure. Reste des sujets d'importance, plus directement liés au problème posé, comme la place des jeunes dans notre société ou la mixité dans le logement social. Malheureusement, c'est là son troisième défaut majeur -est fortement teinté de l'idéologie du « toujours plus de droits individuels » et d'une suspicion généralisée à l'égard de tous ceux qui détiennent une parcelle d'autorité ou de pouvoir. Mais peut-être faut-il ne voir là que l'ultime tentative de recoller les morceaux d'une majorité éclatée ... On connaissait les hésitations et les volte-face du Président de la République sur le plan économique, qui ont tant perturbé certains ; on prend maintenant la mesure de sa ligne sur le plan sociétal : c'est celle de l'émancipation de l'individu sans véritable contrepartie, avec son inéluctable conséquence, à savoir l'effritement de la cohésion sociale ! Ainsi, ce que vous appelez « égalité réelle », notion dont on aimerait d'ailleurs avoir une définition précise, se réduit souvent à une juxtaposition de droits spécifiques en faveur de tel ou tel groupe ou répondant à des demandes particulières de, comme lorsqu'il est proposé d'inscrire la notion d'identité de genre dans notre droit pénal

Un voile de suspicion est également jeté sur nombre de symboles de l'autorité, forcément suspectés d'opprimer ou de freiner l'émancipation des individus, et dont on ne voit pas qu'ils participent aussi, de manière essentielle, à la construction de ces Un nouveau discrédit est ainsi porté aux représentants de l'ordre par des mesures faisant de ceux qui ont la charge de notre protection des suspects. Pour attester de leur probité, les services de police devraient filmer leurs interventions lors de chaque contrôle d'identité. L'État s'autorise à s'immiscer un peu plus dans la sphère familiale, empiétant encore sur la liberté des parents en matière d'autorité parentale. Et vous voudriez réduire encore cette autorité en conférant de nouvelles capacités d'ordre juridique aux mineurs de seize ans, évidemment sans débattre des conséquences en termes de responsabilité Cette défiance à l'égard de toute forme d'autorité va jusqu'à contester l'incarnation même de la démocratie représentative, à savoir les maires, qui voient leur légitimité remise en cause par les prérogatives données aux conseils citoyens, notamment leur capacité d'interpellation du préfet. En matière d'attribution de logements sociaux,

effraie déjà tous les acteurs. À la clef, bien sûr, les sanctions pleuvent, privant les uns et les autres de leurs droits d'attribution pourtant souvent très chers payés ! Quant au fameux article 55 de la loi SRU,

: les communes carencées aujourd'hui sont un peu plus de 200 sur 1 100 communes soumises à l'article 55 de la loi SRU. Avec les objectifs de Mme Duflot, plus de la moitié des communes iront dans le mur pour la prochaine période triennale, et vous faites semblant de ne pas vous en apercevoir. Vous vous enfermez dans une logique absurde de matraquage des communes, qui finira, madame la ministre, je vous le dis parce que je me considère comme un maire bâtisseur, par dégoûter les élus de bonne volonté de faire quoi que ce soit de plus Eh bien, pour nous, à l'impossible nul ne devrait être tenu ; c'est pourquoi, à votre logique du bâton, nous allons substituer celle du contrat entre l'État et la commune. Sur la base d'un constat partagé,

on ne peut qu'être frappé de la vision qui est développée s'agissant de l'avenir professionnel des jeunes. Après les emplois d'avenir subventionnés, votre projet prône le « tout associatif », ce qui consiste en réalité à élargir l'accès des jeunes à une fonction publique ou parapublique déjà pléthorique.

Au-delà des articles, pris un par un, c'est donc la conception même de l'égalité et surtout de la citoyenneté proposée par ce texte qui nous pose problème. La bonne conscience et la candeur avec laquelle vous croyez changer le monde nous semblent aux antipodes des besoins de cette jeunesse en quête d'un destin collectif et surtout de repères. En les gommant toujours plus, vous laissez dans les interstices un vide propice au développement de toutes les idéologies de remplacement. Votre propension à penser une société hors-sol, fondée sur une conception purement théorique de la liberté et une vision désincarnée de la citoyenneté marque une distance toujours plus grande avec le réel. Ce n'est certainement pas de cette manière-là que nous ramènerons dans son giron « les enfants de ces territoires perdus de la République

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, dans le cadre de l'examen en séance publique du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, je souhaite pour ma part attirer votre attention sur le titre II, consacré au logement social, plus particulièrement sur l'article 20, qui vise à réviser et à encadrer considérablement les règles d'attribution des logements sociaux, et ce au nom de la mixité sociale. En effet, cet article prévoit entre autres que tous les bailleurs sociaux devront consacrer au moins 25 % des attributions de logements situés en dehors des QPV au quartile des demandeurs les plus pauvres et, à l'inverse, fixer un objectif d'attribution dans les quartiers les plus en difficulté aux demandeurs plus aisés. Il prévoit également de rendre publics, d'ici à 2022, les critères d'attribution comme les données sur les immeubles et les logements vacants. Il encourage enfin la « location choisie », permettant au demandeur de faire des demandes spécifiques pour les logements qui l'intéressent le plus. Mes chers collègues, je me pose une question simple ces mesures seraient-elles de nature à résoudre les problèmes de mixité sociale ? Je pense très franchement que non qu'elles seraient contre-productives. Grâce à mon expérience en la matière, je connais l'engagement et le dévouement des maires et des bailleurs sociaux. Il ne sert à rien de passer d'une politique de la carotte et du bâton à une politique du bâton et du bâton. Le texte du Gouvernement multiplie les nouveaux critères de priorité pour l'attribution des logements sociaux. Avec une telle multiplicité de priorités, y a-t-il encore des priorités ? Le rôle du Gouvernement n'est pas d'organiser le concours Lépine de la meilleure ou de la moins mauvaise priorité. Nous savons bien que trop de priorités tue la priorité Quelles sont les missions des organismes d'HLM ? Assurer la mixité sociale et loger nos concitoyens les plus modestes. Pourquoi alors intégrer dans le droit commun les personnes relevant du droit opposable au logement, qui doit rester une voie de recours exceptionnelle ? Pourquoi loger prioritairement des personnes qui, si elles sont en situation d'expulsion, ne sont pas dans la légalité ? Cette prime à la mauvaise foi pose d'ailleurs un sérieux problème de principe Pourquoi demander aux bailleurs sociaux de loger prioritairement les personnes connaissant un cumul de difficultés financières et d'insertion ? Nous le savons, l'insertion est une compétence relevant principalement de l'État. doit l'assumer au travers de ses centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dans lesquels le public le plus en difficulté doit pouvoir bénéficier de l'accompagnement de professionnels de l'insertion. Avec ce texte, le Gouvernement fait entrer le logement social dans une logique de quotas. Où est la confiance ? Où est l'autonomie des acteurs de terrain ? Ce sont les élus locaux les organismes d'HLM, avec leur connaissance des spécificités locales, qui sont en mesure d'assurer une politique de peuplement efficace et équilibrée. Comment pouvez-vous croire, madame la ministre, monsieur le ministre, que vous serez plus efficaces dans vos ministères parisiens que ces acteurs de proximité ? C'est, au pire, un péché d'orgueil, au mieux, le témoignage d'une certaine méconnaissance de la réalité de la gestion opérationnelle des bailleurs sociaux. À trop les occuper à à devoir remplir des cases, vous allez les détourner de l'essentiel. Comment espérer, d'ailleurs, qu'ils puissent ainsi sereinement s'atteler à la construction de nouveaux logements, alors que, vous le savez, nous ne construisons pas suffisamment Concernant la question des attributions, le Sénat a redonné de l'oxygène à ce texte. Je remercie Mme la rapporteur Dominique Estrosi Sassone de son travail, de sa disponibilité et de son écoute sur ce sujet. Nous ne sommes pas dupes : avec un tel contrôle des attributions, ce texte participe au final de la tentative de nationalisation de la politique du logement par l'État, au mépris des réalités locales et des élus locaux. Voilà, mes chers collègues, l'essentiel de ce que je souhaitais vous dire en quatre minutes à l'occasion de cette discussion générale. Je laisserai ma collègue Valérie Létard s'exprimer au nom du groupe UDI-UC au sujet des modifications apportées par le Sénat à l'article 55 de la loi SRU. Je conclurai Je conclurai mon intervention par un appel. Le logement social mérite un vrai débat national. Il mérite bien plus que quelques chapitres au sein d'un projet de loi de réconciliation de la gauche, à huit mois de l'élection présidentielle ! La parole est à M.

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, à plusieurs occasions le Président de la République a déclaré que la France avait un grand besoin de simplification. Dans une étude publiée le 27 septembre dernier, comme Mme la rapporteur l'a rappelé, le Conseil d'État s'est alarmé de notre « logorrhée législative », qui « est un enjeu de compétitivité » et « l'un des premiers facteurs d'exclusion » ajoutant que les lois sont souvent prises « en réaction au journal de vingt heures ». Ce texte, après d'autres, est un parfait modèle de cette logorrhée. Au détour de ses 217 articles, le texte issu de l'Assemblée nationale et soumis à la procédure accélérée comporte en effet des dispositions très hétéroclites, touchant au logement, aux gens du voyage, au service civique, en passant par le bizutage, la portabilité du lundi de Pentecôte, la représentation des classes d'âge au sein du CESER, la définition légale des auberges de jeunesse, les conditions de nationalité pour les chirurgiens-dentistes et les débitants de boisson et, pour finir, par l'abrogation d'une ordonnance de Charles X. Cette dernière, je n'en doute pas, est certainement aujourd'hui la première préoccupation de nos compatriotes Ce texte, si vous me permettez l'expression, est un véritable « vide-grenier »- cette opération que l'on effectue lorsque l'on quitte sa maison ou lorsque le propriétaire décide de mettre fin au bail. Pris par le temps, on empile pêle-mêle dans les cartons les bijoux de famille, l'argenterie et la pacotille, au risque d'endommager ou de ne pas retrouver l'important au profit du détail.

sous couvert de lutte contre la radicalisation, remettent en cause une liberté constitutionnelle : la liberté d'enseignement, que l'instruction ait lieu dans la famille ou dans un établissement privé. L'arsenal juridique permettant de lutter contre ces risques existe pourtant, notamment la loi Royal de 1998. J'y reviendrai lors de la discussion de ces articles. Deuxièmement, l'article 47, qui concerne la restauration scolaire, rend obligatoire une compétence facultative des communes, des EPCI, sans même avoir effectué la moindre étude d'impact, et ce à l'heure où les dotations de l'État envers les collectivités ne cessent de diminuer. L'absence d'études d'impact fait d'ailleurs partie des remarques formulées par le Conseil d'État. Le Sénat, à la demande de Françoise Laborde et de moi-même, a rejeté à une très large majorité cette proposition lors de la discussion du texte. Ce projet de loi, comme nombre de textes précédents, démontre la volonté du Gouvernement, mais aussi de sa majorité à l'Assemblée nationale, de tout normer et de tout encadrer. Je veux donc remercier et féliciter nos deux rapporteurs, Françoise Gatel et Dominique Estrosi Sassone, d'apporter un peu de cohérence et de lisibilité en effectuant un tri salutaire. Ainsi, 117 amendements sur les 648 déposés ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 41 ou de l'article 45

entre les déclarations du Président de la République, prônant la simplification, et la réalité à laquelle il est confronté : celle de satisfaire peu ou prou sa majorité composite, qui le contraint à faire l'inverse Ce texte est également révélateur de la volonté du Gouvernement et de sa majorité à l'Assemblée nationale de vouloir tout régler par la loi, donc d'y faire figurer ce qui relève du décret, voire de la circulaire ou du règlement, ajoutant ainsi de la complexité à la complexité. Certes la loi doit être la même partout et pour tous. Toutefois, si la France est une et indivisible, elle n'est pas uniforme. Le respect de cette diversité relève davantage du contrat que que de la contrainte. C'est d'ailleurs le sens des propositions de nos deux rapporteurs. Je les en remercie, d'autant plus qu'elles ont effectué ce travail dans un temps particulièrement contraint. J'associe à ces remerciements le président de la commission spéciale, Jean-Claude Lenoir. Le groupe Les Républicains leur apportera son soutien.

Nous le savons, en politique, il y a des totems et des tabous. L'article 29, qui vise à renforcer une fois de plus les modalités d'application de l'article 55 de la loi SRU fait sans conteste partie de ces symboles qui constituent de véritables marqueurs, suscitant toujours des discussions denses et passionnées. Lors du débat sur la loi du 18 janvier 2013, le Gouvernement a franchi un cap supplémentaire dans le durcissement de cette loi. Nombre d'entre nous avaient souligné les risques d'un élargissement excessif du champ d'application, du passage du taux à 25 %, des conséquences du renchérissement des pénalités et de l'impraticabilité d'une date butoir en 2025. Quand le Gouvernement souhaite raidir encore les choses trois ans après, cela tient un peu de l'acharnement ! Ma position est claire

il a permis la construction de 480 000 logements locatifs sociaux en quinze ans. À part une poignée de communes vraiment récalcitrantes, les autres se sont toutes mobilisées et ont fait des efforts importants de production de logements sociaux. Tout à fait ! Donc, oui, ce dispositif est utile, mais il n'a pas besoin d'être punitif à l'excès. C'est pourtant ce qu'il est devenu au fil du temps et des textes, ce qui le rend trop souvent impossible à mettre en oeuvre. C'est la raison pour laquelle

! La contractualisation, comme je l'ai souligné et comme l'a montré Dominique Estrosi Sassone, doit permettre de redonner à ce dispositif toute la souplesse nécessaire, mais nous devons dans le même temps conserver l'objectif initial de la loi, qui est bien la construction de logements locatifs sociaux là où les besoins s'en font sentir. Or la loi de 2013 a multiplié les contraintes, au risque de démobiliser les meilleures bonnes volontés. Eh oui ! Le résultat, c'est le constat établi par le deuxième rapport du CGEDD sur l'application de l'article 55. L'objectif de 25 % de logements sociaux en 2025 sera impossible à tenir pour de très nombreuses communes. Il faut donc revenir à la raison. Néanmoins, devons-nous pour autant abandonner tout cadrage et laisser à la contractualisation la liberté de tout fixer ?

et en l'inscrivant dans le dispositif proposé par la commission spéciale et Mme la rapporteur, il me semble possible d'adopter une voie médiane, qui « décorsète » l'article 55- il en a besoin -sans le dénaturer. C'est d'ailleurs l'objet des principaux amendements que j'ai déposés, avec le soutien d'un grand nombre de mes collègues du groupe UDI-UC. Ces amendements visent notamment la question des catégories de logement assimilées à du logement social : où est-il pertinent de placer le curseur ? Ils ont également pour objet la détermination du taux de logements locatifs sociaux.

Je rappelle que les organismes de logements sociaux municipaux seront transférés à l'intercommunalité dès 2017 et que les EPCI sont, au travers des PLH, le lieu de programmation et de contractualisation des politiques locales de l'habitat.

Ne faisons pas de l'article L. 302-5 une coquille qui ne serait pas assez remplie quand des besoins nombreux existent encore. Ne stoppons pas l'effort aujourd'hui, ce qui reviendrait à en exonérer les communes qui ont été les moins vertueuses ! Ne passons pas d'un excès à l'autre. En même temps, gardons à l'esprit que la mixité sociale ne se décrète pas ; cela se construit en s'inscrivant dans des stratégies locales englobant non seulement le logement et l'accompagnement social, mais aussi l'économie, les transports et les services aux populations. Soyons justes et équitables. Faisons confiance aux collectivités

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, sur ce projet de loi, l'Assemblée

principe d'ardente obligation de la Nation tout entière de permettre la réalisation d'un engagement citoyen », « République en actes », « égalité réelle

que le meilleur moyen de les promouvoir soit de les invoquer sous forme incantatoire pour habiller des dispositions qui, par leur caractère irréaliste et caricatural, les discréditent. Ces incantations signent un aveu d'impuissance. Que peut par exemple signifier « l'égalité réelle », qui supposerait l'existence fumeuse d'une « égalité irréelle »

troisième défaut est cette obsession de vouloir tout sanctionner, verrouiller, imposer, uniformiser, au mépris des réalités du terrain, et au profit d'une vision autoritaire et moralisante de l'action publique, exercée par un État centralisateur. Renforcer les sanctions infligées aux communes carencées, élargir les prérogatives des EPCI et du préfet par substitution aux maires, autant de mesures manquant de pragmatisme au nom de l'idéologie. conséquence, de nombreuses mesures sont, en l'état, inapplicables. D'où le recours aux ordonnances, pourtant violemment critiqué en 2005 par un député devenu depuis lors Président de la République,

à la procédure d'urgence ... Le quatrième défaut est que l'État légifère et envoie la facture à d'autres, en l'occurrence aux collectivités territoriales dans un contexte de baisse des dotations. Bien sûr ! En un mot, il s'agit d'une loi de recentralisation, aux antipodes des affirmations de décentralisation et de simplification. Finalement, ce projet de loi constitue à lui seul le résumé d'un quinquennat pour rien, placé sous le signe des contradictions, où le verbiage l'emporte sur le pragmatisme. ce texte n'a-t-il pas d'autre objet, après le pathétique feuilleton de la loi El Khomri, qui a cruellement mis en lumière les divisions profondes de la majorité à l'Assemblée nationale, que de chercher à rassembler ce qui reste de la majorité et de séduire un électorat qui déserte. déserte. Je veux rendre hommage au travail de la commission spéciale, qui s'est efforcée de donner un cadre juridique à ce texte relevant plus du déclamatoire que du législatif. Je salue tout particulièrement le travail de nos deux rapporteurs.

qui a été accepté par la commission spéciale, sur la dégressivité des indemnités pour les fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Cet amendement n'a absolument rien à voir avec le texte,

Nous vous avons accompagné dans la réforme du règlement du Sénat. Nous soutenons votre volonté d'être plus efficace et de passer moins de temps sur les textes. Néanmoins, ce travail de clarification ne peut devenir un prétexte, dans le contexte préélectoral que nous connaissons tous,

acte vous est donné de votre rappel au règlement. À la demande du président du Sénat, je voudrais vous faire la réponse suivante.

Le droit d'amendement est un droit fondamental, qui doit s'exercer dans les conditions fixées par la Constitution. Nous avons tous constaté, ces dernières années, une hausse continue du nombre d'amendements- jusqu'à 10 000 lors d'une précédente session -, ce qui pèse sur l'organisation de notre temps parlementaire et crée de l'inflation législative. Le projet de loi que nous allons examiner est passé à l'Assemblée nationale de 41 à 217 articles. Il a donc connu un quintuplement du nombre de ses articles fou ! Conformément aux recommandations du groupe de réflexion sur les méthodes de travail, le bureau du Sénat et la conférence des présidents ont préconisé, le 11 mars 2015, que les irrecevabilités constitutionnelles soient mises en oeuvre dans le respect du droit d'amendement, qu'il s'agisse des articles 40, 41 ou 45 de la Constitution. À nous de faire confiance au travail des commissions, en l'espèce celui de notre commission spéciale et de ses deux rapporteurs, sous la conduite de son président, Jean-Claude Lenoir. Il y va de la qualité de notre travail

remercier l'ensemble des membres de la commission spéciale qui ont travaillé sur ce texte. J'avais averti les candidats à cette fonction que ce travail serait mené

recours massif aux automates ... Nous assistons à une accélération de la réduction du réseau postal, et cela en tout point du territoire. C'est vrai ! Cette offensive se traduit aussi par la précarisation de l'emploi et par des techniques managériales fragilisant les personnels.

des besoins de proximité et l'exigence de qualité de service pour tous, habitants comme acteurs économiques. Pourtant, ces missions de service public sont aujourd'hui directement menacées par des logiques de rentabilité financière de court terme. En effet, au nom de l'adaptation du réseau aux contraintes économiques, la fermeture de très nombreux bureaux de poste s'accélère dans le monde rural et concerne maintenant les villes. La Poste passerait ainsi d'un réseau où les bureaux de poste étaient largement majoritaires à un réseau tout à fait dominé par les partenariats, où leur nombre serait en forte régression. alors que le contrat de présence postale territoriale pour les trois ans à venir est en cours de discussion, que va faire l'État actionnaire pour mettre un terme à la fermeture de ces bureaux ?

vous avez raison : la présence postale est indispensable à une politique harmonieuse d'aménagement du territoire. C'est l'un des services publics les plus importants pour les Français, même si le statut de La Poste a évolué. Je suis bien naturellement

Il permettra de maintenir et de moderniser les 17 000 points de contact existant, pour tenir compte de l'évolution des usages. Il financera également une partie des 500 maisons de services au public

La Dépakine, médicament antiépileptique, est aujourd'hui au coeur d'un véritable scandale sanitaire. Ses effets tératogènes, qui provoquent des malformations chez le foetus, sont mentionnés dans de nombreuses études scientifiques, et cela depuis 1982.

de loi que j'ai déposée le 25 février dernier. Elles réclament également la mise en oeuvre d'un fonds d'indemnisation. Au début de nos échanges, vous étiez plutôt opposée à l'idée d'un pictogramme. Finalement, et je m'en félicite, vous en acceptez le principe et je crois savoir que les choses évoluent

Il est en effet capital que la firme pharmaceutique ne puisse pas le modifier au gré de ses envies. Des faits graves de conflits d'intérêts entre l'ANSM et certains laboratoires ont déjà été mis au jour dans le passé. N'oublions pas les missions de cet organisme : autoriser, surveiller, contrôler et informer ! Nous avons la chance de posséder un organisme public, le Centre de référence sur les agents tératogènes, le CRAT, qui dresse la liste de l'ensemble des molécules à risques. arrêté, le logo que les familles réclament sur l'ensemble de ces molécules permet d'éviter des récidives. C'est un geste préventif ! L'État et le laboratoire doivent prendre leurs responsabilités au sein de cette affaire, afin d'indemniser au mieux les familles. Aussi, madame la ministre, quand comptez-vous prendre les mesures qui s'imposent pour répondre pleinement aux attentes et pour éviter de nouveaux problèmes ? La parole

de la Dépakine soient justement et rapidement indemnisées. Je le dis sans difficulté et sans ambages, la Dépakine est un médicament

appelant l'attention des personnes qui prennent de la Dépakine ou d'autres médicaments du même type sur les risques en cas de grossesse. Vous le voyez, monsieur le sénateur, j'avance, avec l'APESAC, dans l'intérêt des victimes, car c'est la seule chose qui retient mon intérêt dans

Monsieur le ministre, le Gouvernement a présenté ce matin des dispositifs visant à soutenir la profession agricole, durement touchée par les effets de marché et les aléas climatiques. Nous prenons acte de ces mesures, et je salue le principe de renégociation des emprunts, ainsi que les efforts proposés sur le foncier non bâti.

de moins de normes ! Or, au moment même où vous annoncez ce plan, se profile de manière contradictoire la réécriture d'un arrêté relatif aux règles environnementales sur l'utilisation des produits l'expression, monsieur le ministre, met le feu aux campagnes ! Cet arrêté, retoqué par le Conseil d'État pour de simples raisons de forme, ferait l'objet d'une réécriture beaucoup plus contraignante sur le fond. non traitées, les ZNT, aux habitations, aux forêts, aux haies, aux bosquets et aux bois, élargissant ces zones de 5 à 20 mètres, voire à 50 mètres. Cela susciterait un recul majeur du chiffre d'affaires des agriculteurs : une première simulation dans mon département des Yvelines indique que plus de 15 000 hectares seraient affectés, soit 16 % de la surface agricole utile. Ce serait une véritable provocation

Monsieur le ministre, nous sommes à la veille de l'ouverture du 86 congrès de l'Assemblée des départements de France, l'ADF, qui va se Hier promis à la disparition sous un faux prétexte d'économie, les départements ont franchi le cap de la loi NOTRe et se sont vus conforter dans leurs missions de solidarités humaines et territoriales. Le département se trouve donc renforcé en tant qu'échelon intermédiaire, dans la proximité avec les communes et les intercommunalités et en lien fort avec les régions. Les élus départementaux ont à coeur de mettre en oeuvre des politiques innovantes, au service de chacun des habitants et pour tous les territoires, urbains et ruraux. Certains parleront aujourd'hui des allocations et du RSA, sujets d'inquiétude pour les départements. Je souhaite, pour ma part, évoquer la mission territoriale de l'assemblée départementale, qui vise au développement équilibré entre ville et campagne. Les travaux engagés avec les préfets et les élus locaux pour un accès facilité aux services publics de qualité concernent l'ensemble de nos territoires, en particulier les plus délaissés d'entre eux. Justement, solidaire avec ces territoires, je veux saluer votre initiative de mise en place des contrats de ruralité, instruments visant à développer les territoires ruraux et à accélérer la réalisation de projets concrets au service des habitants et des entreprises. Ma question est donc simple : quelle place souhaitez-vous réserver aux départements dans les contrats de ruralité, pour accompagner au mieux communes et intercommunalités rurales face aux difficultés du quotidien ?

la sénatrice, de souligner l'importance des départements dans le cadre des politiques de proximité et leur rôle indispensable dans l'organisation institutionnelle de la France. Je crois d'ailleurs avoir démontré en mon temps mon attachement personnel

par souci d'équité et de complémentarité entre territoires urbains et ruraux, de créer les contrats de ruralité, qui sont en quelque sorte les pendants des contrats de ville ; de déconcentrer auprès des préfets, toujours dans une volonté de proximité ;

Et l'on ne parle ici que des véhicules homologués depuis 2009, mais dont les tests ont été faits en laboratoire et qui sont classés Euro 5 et Euro 6. Il faudrait donc leur ajouter des millions de véhicules plus anciens. Malheureusement, nos constructeurs nationaux

que les personnes qui ont été incitées à acheter du diesel pendant des années seraient aidées à remplacer leurs véhicules par des modèles moins polluants. Vous avez également annoncé des bonus renforcés pour les véhicules électriques. C'est une bonne chose. Nous regrettons toutefois l'abandon apparent de l'évolution de la TVA sur les carburants, qui supprimerait l'avantage compétitif de l'achat de véhicules diesel par les entreprises. Nous attendons surtout, au-delà de ces annonces, des décisions concrètes. Madame la secrétaire d'État, ma question est simple. Que fait-on de ces millions de véhicules bien trop polluants ? Quel plan global allez-vous mettre en oeuvre, au vu de l'urgence de la situation sanitaire ? Comptez-vous mettre en place des rappels de véhicules ou des compensations pour les propriétaires de ces voitures ? La parole

13 recommandations ont été proposées. La dernière réunion de la commission indépendante s'est tenue le 22 septembre dernier. Il a été décidé qu'elle poursuivrait ses travaux sur la base de nouveaux essais, réalisés au sein de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Dans les cas où des dysfonctionnements ont été constatés, des plans d'amélioration pour les nouveaux véhicules produits, ainsi que pour les véhicules déjà en circulation, ont été mis en place. Le ministère vérifiera que les améliorations sont efficaces en termes de dépollution. Cette situation doit nous engager à nous tourner résolument vers le transport propre. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017 et des investissements d'avenir, des mesures ont été prises : pour les particuliers, le bonus-malus et la prime à la conversion, destinés à accélérer la transition vers les véhicules propres, ou le crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge pour les entreprises, le relèvement du plafond d'amortissement des véhicules à faible émission de 18 300 à 30 000 euros ; pour les collectivités locales et l'État, les prêts pour la croissance verte de la Caisse des dépôts et consignations aux collectivités locales, soit 5 milliards d'euros destinés au financement des territoires à énergie positive.

Alep, « ville martyre », sous un déluge de feu : un hôpital détruit par des armes anti-bunker ; l'utilisation d'armes chimiques et de barils de chlore Il y a encore 300 000 survivants et 100 000 enfants affamés et enfermés. On ne sort pas d'Alep ! Alep est « au coeur de la tragédie syrienne Au-delà des mots « barbarie » et « crime de guerre », la trêve est rompue et les Occidentaux ne réagissent pas. Les ruines d'Alep sont aussi celles de la conscience internationale. Au-delà du discours du président Hollande à l'ONU- la France avait raison en 2013 ! -, au-delà du silence d'Obama et des États-Unis « à bout de patience », tout est-il bloqué ? Comment mobiliser autour de la France la communauté internationale ? Quelle pression morale peut-on exercer, ou espérer, pour répondre aux cris des Syriens et sauver des vies à Alep ? Comment gérer la stratégie russe, celle de Poutine, maître du jeu au Moyen-Orient soutenant le régime implacable de Bachar, et peut-être son maintien au pouvoir ? Comment éviter l'impasse avec la Russie ? Est-ce le retour à la logique des

aujourd'hui en Syrie, est de tout faire pour mettre fin au déluge de violence qui submerge Alep depuis maintenant une semaine. Vous avez rappelé, avec précision et force, l'horreur des exactions qui se déroulent dans cette ville aujourd'hui martyre. Ce qui se passe à Alep, cette logique de guerre totale, est sans précédent, y compris dans ce conflit qui, pourtant, n'a pas été avare d'horreurs. Ce déchaînement de violence, qui cible les civils, en particulier les hôpitaux et les personnels de santé, est monstrueux et inacceptable. Ce sont des actes constitutifs de crimes de guerre, et leurs auteurs devront en répondre, y compris devant la justice internationale. Comment y mettre un coup d'arrêt ? Certains préconisent un alignement total sur Moscou au nom de la lutte contre le terrorisme. D'autres, à l'inverse, estiment que nous devons rompre avec Moscou. Soyons clairs, et le ministre des affaires étrangères l'a indiqué sans ambiguïté, aucune de ces deux options ne permettra de mettre fin au drame qui se déroule sous nos yeux. Il y a deux pistes d'action. La première est la voie diplomatique. La France travaille en ce sens au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, où nous sommes engagés dans la négociation d'une résolution, afin d'établir un cessez-le-feu et de permettre aux populations civiles d'Alep de recevoir une aide humanitaire. Cette négociation est compliquée, mais elle se poursuit. Le moment de vérité approche, et la France prend toute sa part dans la négociation, comme il se doit, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. La seconde piste d'action est le volet humanitaire. L'Union européenne a lancé une initiative, en lien avec les Nations unies, pour que l'aide humanitaire soit acheminée sans délai et que les blessés puissent être évacués. La France, là aussi, prend toute sa part, et nous sommes en contact étroit avec Mme Federica Mogherini, avec un seul objectif : mettre fin au martyre d'Alep.

multiplie les déclarations et les discours à sa propre gloire, qui vont de « J'ai redressé les comptes de la sécurité sociale » à « J'ai sauvé la sécurité sociale » ! La Cour des comptes est moins laudative ... Elle relève un déficit en 2015 moindre que prévu, mais toujours élevé, encore supérieur à celui de l'avant-crise, une trajectoire de retour à l'équilibre incertaine, avec une dette sociale inquiétante. Qui plus est, même la Commission des comptes de la sécurité sociale prévoit un déficit situé entre 9,1 et 9,8 milliards d'euros. Facétieux, M. le ministre Sapin, dans sa communication du 25 mars dernier, annonçait triomphalement que « la dette de l'État a connu en 2015 sa plus faible progression depuis 2007 Or, le même jour, la Cour des comptes formulait une réserve dans son rapport annuel sur les chiffres de la dette et dénonçait un arrangement comptable pour camoufler soigneusement le gonflement de ladite dette, qui est aujourd'hui de 2 710 milliards communication de Mme Vallaud-Belkacem, qui, lundi, renvoyait le pape à la relecture de nos livres scolaires. Elle devrait elle-même s'y pencher : les cours en lien en lien avec la théorie du genre actuellement dispensés au collège s'appellent « les cours sur l'identité en construction ». Il faut bien reconnaître, mes chers collègues, que, avec les programmes scolaires de Mme Vallaud-Belkacem, c'est la France qui prend congé d'elle-même communication de M. Eckert, secrétaire d'État au budget, qui « assure que le Gouvernement aura effacé l'année prochaine l'ensemble des hausses d'impôts et taxes sur les entreprises ». Pour ce faire, il ne manque que 16 milliards d'euros ! Insondable est la communication de M. le ministre de la recherche : deux décrets d'avance lui rabotent par centaines

saluer le travail de la ministre des affaires sociales, qui a su au fil de ces années, sans aucun déremboursement et en maintenant la protection sociale de tous nos concitoyens, rétablir

Madame la ministre, l'hôpital était il y a quelques années encore un sanctuaire républicain, un lieu d'accueil ouvert aux souffrances et aux détresses humaines. Or, en quelques années, on a vu s'y développer une violence à laquelle les personnels hospitaliers sont quotidiennement confrontés. En témoigne l'instauration d'un Observatoire national des violences en milieu de santé, l'ONVS, dont le récent rapport fait état de 14 502 atteintes aux personnes et aux biens pour l'année 2014, touchant ainsi plus de 18 000 personnes Patients et accompagnants sont hélas à l'origine de l'essentiel de ces actes de violence, généralement liés à leur prise en charge, au temps d'attente, à l'absorption d'alcool ou de stupéfiants. Un acte de violence intervient en moyenne toutes les 30 minutes, accompagné d'injures, d'insultes et de provocations. Ces actes traduisent la banalisation de la violence, elle-même témoin du délitement des moeurs dans notre pays. Je tiens tout d'abord à rendre hommage au personnel hospitalier, dont le travail est déjà difficile et qui subit avec sang-froid et dignité cette évolution que vous semblez croire inéluctable. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour mettre un terme à ces dérives inadmissibles ? Ne pensez-vous pas que cette escalade et sa banalisation sont le reflet d'une société minée par la culture de l'excuse ?

nous avons décidé que les hôpitaux les plus exposés seraient désormais intégrés dans les circuits de patrouille mobile Vigipirate et Sentinelle, car, à côté des violences du quotidien, existe aussi le risque de violence terroriste, que nous devons prendre en considération. Par ailleurs, chaque établissement devra élaborer un plan de sécurité intérieure. Des financements seront apportés progressivement : un plan de 75 millions d'euros sur trois ans sera mis en place à partir de 2017. Ces place à partir de 2017. Ces financements nécessaires bénéficieront, d'abord, aux établissements prioritaires. Vous le voyez, monsieur le sénateur, nous ne nous résignons pas face à la violence : nous dégageons des moyens et nous mettons en place une politique active et volontariste.

songe à panser les plaies, mais jamais à soigner les causes. On ne réglera la question qu'avec une réponse globale. Or, aujourd'hui, deux chiffres clefs se contredisent : l'augmentation des actes de violence et la hausse des classements sans suite des plaintes déposées par les hôpitaux. Vous vous contentez de poser des compresses sur une société que vous contribuez à rendre malade. La parole est à Mme Nelly Tocqueville, pour le groupe socialiste et républicain. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement. Les agriculteurs traversent des crises successives depuis plusieurs années. Les récentes évolutions du prix du lait et de la viande en sont des témoignages douloureux. Certaines de ces crises sont structurelles et appellent des réponses à long terme, pour faire évoluer notre modèle agricole. D'autres sont plus conjoncturelles ou sanitaires, notamment dues aux conditions climatiques. Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous avez reçu les représentants des organisations professionnelles, avec lesquels vous avez évoqué les difficultés rencontrées par un certain nombre d'exploitants, faisant suite, en particulier, aux médiocres moissons de céréales en 2016, comme c'est le cas dans mon département, la Seine-Maritime, ou encore dans le Poitou et le bassin parisien. Au niveau national, avec 29 millions de tonnes de grain annoncées, cette année sera celle de la plus faible récolte depuis 1986, la baisse atteignant parfois Au reste, cela risque fort d'avoir un effet sur nos exportations et, par contrecoup, sur l'activité du Grand port maritime de Rouen, premier port céréalier européen. À ces difficultés s'ajoute une baisse des prix, du fait des bonnes récoltes enregistrées, sur le plan tant de la qualité que de la quantité, à l'échelle mondiale. Ainsi, la faiblesse de la production nationale, la qualité médiocre du grain et des prix bas peuvent avoir des conséquences irréversibles pour certaines exploitations, déjà fragilisées, particulièrement celles de polyculture d'élevage, d'autant plus quand elles doivent assumer des remboursements de mise aux normes ou des investissements en matériel. Enfin, les exploitants s'inquiètent du blocage du dispositif de modulation des aides attribuées au titre de la Monsieur le ministre, vous avez annoncé ce matin un plan d'aide, volontariste et fort, pour soutenir ces exploitations en difficulté. Ce plan fait suite aux dispositifs européens sur le lait que vous avez obtenus en 2015 et 2016.

quand notre dette dépasse les 2 000 milliards d'euros et les 100 % du PIB, sans que cette dépense publique fasse de notre pays un paradis, je me dis qu'il y a un problème. Aussi, en écoutant les promesses de campagne des uns et des autres, je m'inquiète : partout, c'est « dépenses à tout va », et Bruxelles redevient le bouc émissaire. Je vous le dis très sincèrement, je n'ai pas envie que la France devienne le Royaume-Uni, la Hongrie ou encore la Pologne. Je n'accepte pas que l'on verse sans arrêt dans l'ou dans l'euroscepticisme. L'Europe de ces dernières années est sans doute médiocre, incompréhensible, bureaucratique et pas assez démocratique. Oui, c'est vrai. elle reste un modèle jamais surpassé de relations entre États démocratiques, qui permet de grandes avancées. Aussi, je souhaite que la France réagisse aux votes intervenus ailleurs en Europe. Il y a un besoin urgent d'Europe. Qu'entendez-vous faire pour y répondre ? Quelle relance européenne la France appelle-t-elle de ses voeux, alors que l'accord de Paris va entrer en vigueur ? La voix de la France est attendue.

quand l'Allemagne était revenue à l'équilibre. Depuis lors, il a été nettement réduit et il repassera sous la barre des 3 % l'année prochaine, pour permettre notamment à la dette publique de se stabiliser, à bonne distance du seuil des 100 % du PIB que vous avez loi de finances pour 2017, le Gouvernement a ainsi confirmé l'objectif de ramener le déficit public à 2,7 % du PIB. Cet engagement, nous le tiendrons ! Nos résultats passés, reconnus et salués

suppression du droit de publication pour les mineurs, suppression de la garantie d'accès aux cantines scolaires, y compris pour les enfants de chômeurs, suppression du droit d'interpellation pour les conseils citoyens. On peut déconstruire,

Monsieur Favier, comment accuser le Gouvernement, contre lequel vous avez eu des mots très forts, de ventiler la pauvreté sans y remédier ? Bien sûr, personne ne nie

l'évolution progressiste vous a toujours été imposée, car vous êtes incapables de faire la moindre proposition en ce sens. Les Français auront l'occasion de juger vos propositions dans quelques mois

d'enseignements contraires aux valeurs de la République. Nous devons nous donner les moyens de prévenir d'éventuels foyers antirépublicains. Vous avez des solutions, nous en avons d'autres. Nous pensons que les nôtres sont plus efficaces. Je ne vois pas ce

particulièrement difficiles, souvent obscures, le combat pour la liberté, auquel nous nous sommes, à un moment de notre histoire, identifiés, puissent recevoir l'appui symbolique et la reconnaissance de la France.

qui, « par leurs écrits et leur courage, ont servi la cause de la liberté ». Or le droit de la nationalité ne doit être modifié que d'une main tremblante- pour reprendre une expression déjà évoquée -, dans un projet de loi spécifique et avec une étude d'impact complète. Certains termes de votre amendement pourraient laisser une trop grande marge de manoeuvre : comment définir ce qu'est un « service exceptionnel » ? Je rappelle que le droit en vigueur prévoit déjà des mesures en ce sens la naturalisation est possible pour les étrangers qui ont « rendu des services exceptionnels à la France ou dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel » ; le nouveau « passeport talent » peut être délivré aux étrangers dont la « renommée nationale ou internationale est établie

prévoit déjà, comme l'a souligné Mme la rapporteur, d'accorder la nationalité française à un étranger qui aurait rendu des services exceptionnels à la France. Le code civil offre cette possibilité, qui est régulièrement utilisée. Dans ce cas, le décret de naturalisation est rendu après avis du Conseil d'État,

de réfugié à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Comme vous le savez, l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié peut être naturalisé sans condition de stage, conformément à l'article 21-19 du code civil. Le régime actuel

Je voudrais insister sur le fait que notre pays, dans ce monde troublé, a besoin d'être vu par l'ensemble des peuples du monde, comme toujours porteur du flambeau de cette lumière. Il est doit être le phare de la liberté.

que la liberté est une petite flamme toujours vacillante qu'il faut entretenir avec beaucoup de vigilance pour qu'elle ne s'éteigne pas. C'est le rôle de la France. Ceux qui se battent pour la liberté font souvent référence à notre pays.

La volonté de fusionner les réserves civiles existantes dans un service civique unique part, me semble-t-il, d'un constat assez éclairé, celui de dispositifs épars et peu complémentaires. je ne suis pas certaine que ce choc de simplification soit suffisant pour régler la situation. Pour ne prendre qu'un exemple, l'instauration de la réserve citoyenne de l'éducation nationale, en janvier 2015, pose question quant à sa réelle efficacité. le nombre d'inscrits est relativement élevé, les réservistes ont été peu mobilisés. L'une des raisons régulièrement invoquées est le manque de coordination entre ces acteurs nouvellement disponibles et les structures, plus anciennes, comme la Ligue de l'enseignement ... N'y ... N'y aurait-il pas là une piste de .travail à approfondir pour permettre une meilleure mobilisation des réservistes, dans les limites du respect des autres formes d'engagement et de celles et ceux qui en font leur métier ?

sur le départ ou déjà partis. Nous espérons, dans ce domaine, que la charte prévue dans cet article contribuera à cadrer efficacement ce dispositif plus qu'intéressant. La parole est à M.

c'est à l'évidence parce que nous sommes confrontés à la multiplication des attentats terroristes. Or il apparaît que la réponse n'est pas du tout à la hauteur du problème.

par des terroristes musulmans, recrutés dans les sphères communautaristes musulmanes. C'est donc contre le communautarisme qu'il faut lutter ; en ce n'est certainement pas en créant une réserve citoyenne que l'on va inciter les terroristes potentiels à rentrer dans le droit chemin. On vise complètement

et qu'elle « n'est efficace que si elle existe partout et en tout temps ». Il poursuivait en précisant que la démocratie « ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire pendant cinq ans. Elle est action continuelle du citoyen. » Cette « action continuelle du citoyen » peut prendre plusieurs formes

d'ailleurs l'objet de ce projet de loi et, singulièrement, de son titre I. Parmi ses principales mesures, on peut citer l'instauration de la réserve civique, la valorisation de l'expérience acquise lors de la réalisation d'un service civique ou encore la volonté de faciliter l'exercice de responsabilités associatives, ce que permettait l'article 8, malheureusement supprimé par la commission spéciale. J'aurais aussi aimé, mes chers collègues, évoquer devant vous des expériences telles que les coopératives jeunesse de services, qui permettent à de jeunes mineurs, à partir de seize ans, de s'engager dans de véritables projets d'éducation et d'entrepreneuriat situés au croisement de la sphère économique et de l'éducation populaire. C'était un amendement d'appel, mais il a été déclaré irrecevable au titre de Depuis les tragiques événements qui nous ont frappés, nombreux sont ceux qui ont ressenti la nécessité de résister et de s'investir, comme en témoigne l'engouement pour la réserve opérationnelle. La solidarité est apparue comme une réponse à la barbarie ; l'engagement, comme un puissant facteur de résilience et de catharsis. La jeunesse a réagi en manifestant son irrémédiable besoin d'agir et son envie d'engagement. Aux « déclinistes » et aux identitaires, elle apporte une réponse concrète et sans équivoque : l'engagement est une valeur partagée qui fonde notre identité collective. Ce qui crée du commun, c'est précisément cet engagement peu importent nos différences ! Très bien ! Toutefois, l'engagement ne se décrète pas. Il ne précède aucunement le sentiment d'appartenance à une collectivité ; au contraire, il en est une émanation. Pour cette raison, les inégalités et les fractures qui nuisent à la cohésion d'une société sont autant de causes qui freinent l'engagement. C'est pourquoi je veux saluer ce projet de loi qui, par son titre I, mais aussi son titre II, consacré à la politique de mixité sociale, va pouvoir en témoigner. En conclusion, mes chers collègues, je crois qu'il faut se souvenir que les bâtisseurs de murs ont toujours épuisé la démocratie, quand les bâtisseurs de ponts l'ont toujours fait vivre

Je soutiens totalement la réserve citoyenne, qui permet l'expression d'une nouvelle forme de patriotisme. Néanmoins, après les belles paroles des rapporteurs et leur érection en victimes de la mauvaise foi des lobbys et de l'opposition sénatoriale, coupables de dénigrer la bonne foi et l'excellent travail du Sénat, je tiens je tiens à exprimer mon désappointement, mon incompréhension, voire mon indignation. Alors que, ces derniers mois, le Sénat avait su se rassembler en faveur d'amendements que j'avais présentés dans différents

Cet amendement visait à introduire dans l'article 1 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations un alinéa prévoyant, dans la formation initiale et continue des professionnels de justice, une formation sur la spécificité de l'accueil et de l'accompagnement des justiciables avec handicap. Cette formation leur permettrait de mieux comprendre le handicap et de mieux le prendre en compte dans l'exercice de leurs missions. En quoi cet amendement déroge-t-il à l'esprit de la loi Égalité et citoyenneté ?

quelle explication allons-nous donner à Droit pluriel, au Défenseur des droits et à toutes les associations représentatives qui constatent, à juste titre, les inégalités d'accès, d'accompagnement et de traitement par la justice de notre pays, qui méconnaît les particularités du handicap ? si le Sénat est sensible à la condition des femmes, il est en revanche insensible à celle des personnes avec handicap ? Attention, chers collègues, la France des porteurs de handicap nous regarde ! Eux-mêmes, leurs familles, leurs amis et leurs défenseurs nous regardent et vous jugeront

commission ? Ma chère collègue, je salue la qualité de votre intervention et je sais que vous avez effectivement eu à coeur

revenir aux fameux six points de notre méthode, mais, dès lors que les choses sont possibles en l'état du droit, nous avons jugé utile de ne pas inscrire dans la loi cette faisabilité. Il ne s'agit pas

ce sujet, selon des critères de réalisme, nous nous interrogeons sur la capacité des consulats, compte tenu de leurs moyens humains et financiers, à assurer le développement du service civique dans les villes où ils sont implantés. Par conséquent, ma chère collègue, vous me voyez navrée- je vais devoir passer la semaine à être navrée et à m'excuser

que la réserve civique « peut comporter des sections territoriales instituées par convention entre l'État et une ou plusieurs collectivités territoriales ». Je ne vois pas pourquoi les Français de l'étranger seraient exclus du bénéfice de cet article, même si,

la réserve citoyenne sur le territoire de pays étrangers, pourquoi alors nos amis algériens ne viendraient-ils pas créer chez nous des sections de la réserve citoyenne algérienne ?

d'un autre État. C'est à la mode maintenant : tout le monde s'occupe de tout, il n'y a plus de citoyenneté, il n'y a plus rien ! Quant à moi, j'ai une conception très stricte de la souveraineté nationale et, de même que je souhaite que la souveraineté nationale de la France soit respectée, je pense qu'il convient que la France respecte celle des autres États.

dans les écoles françaises, dans les alliances, là où ils sont utiles. Créer la réserve civique des Français de l'étranger ne revient pas à constituer des milices à l'étranger ! La parole

tant les 150 000 emplois supprimés par la RGPP ont mis à mal les services publics. De fait, certaines communes pourraient être tentées d'avoir recours à des réservistes pour des opérations que des agents publics auraient pu ou dû effectuer. Par ailleurs, il se pourrait aussi que des collectivités, voire l'État lui-même, fassent l'économie d'un recrutement de fonctionnaires au profit du recours aux réservistes. C'est pour éviter cet effet pervers que nous avons déposé cet amendement. Il nous semble que nous sommes là face à un sujet qui mérite de la prudence de la part des parlementaires. C'est pourquoi nous proposons que soit inscrit dans la loi le principe de non-substitution, comme pour le service civique. La parole

Françoise Laborde. Le présent amendement vise à rétablir la désignation d'un tuteur pour les réservistes mineurs, obligation qui n'est pas, selon moi, très contraignante pour la structure d'accueil. En effet, l'article 1 est clair : « La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel,

auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l'article 1, aux règles de service de l'organisme. » Je pense donc qu'un mineur peut être accompagné dans son apprentissage et sa connaissance des valeurs républicaines. Quel

mais qui n'ont pas besoin de les former de manière trop rigoureuse. Je demande de la souplesse et de l'efficacité. Tel est l'esprit de la réserve civique : faire face à un besoin immédiat et urgent dans des conditions d'efficacité qui ne doivent pas être alourdies par le tutorat proposé par Mme Laborde. L'avis du

soient, par cet article, pleinement associés à la réserve civique. On donne ainsi une très bonne nouvelle au 1,7 million de Français qui vivent à l'étranger et qui, bien qu'ils soient éloignés géographiquement de notre pays, y restent profondément attachés.

Nombre d'entre eux agissent pour faire vivre la communauté française au quotidien. Certains s'engagent bénévolement dans des associations, d'autres organisent des débats sur la vie politique ou culturelle française. Je le répète, Je suis convaincue, mes chers collègues, qu'utilisée avec intelligence, et elle le sera, la réserve civique permettra de renforcer la vitalité des forces vives françaises de l'étranger. Il ne fait aucun doute que de nombreux compatriotes souhaitant servir l'intérêt général se manifesteront auprès des postes consulaires, qui pourront, selon les missions ou les besoins, les répartir auprès des lycées et instituts français,

parmi les Français établis hors de France afin de constituer la réserve civique à l'étranger

que l'ensemble des réserves citoyennes composant la réserve civique étaient ouvertes aux Français de l'étranger, dans les mêmes conditions qu'en France, alors que certaines réserves, notamment la réserve citoyenne de la police nationale, ne pouvaient être adaptées hors du territoire national

dans l'Hexagone, alors que, pour les dispositifs de réserve citoyenne à l'étranger, par respect pour la souveraineté des pays d'accueil, les réservistes ne peuvent être que de nationalité française. Cet amendement vise donc à favoriser le développement des réserves citoyennes à l'étranger en les dotant d'une base juridique solide. Il ne crée pas de charge budgétaire nouvelle, ces réseaux existant déjà à l'état embryonnaire et leur animation pouvant être confiée à des associations comme l'Association internationale des réservistes citoyens, en lien avec les attachés de défense et conseillers consulaires.

-tenir compte de cette nouvelle responsabilité pour adapter ses moyens aux demandes éventuelles. Laisser cette organisation libre permet à chaque poste diplomatique, dans le respect des principes généraux de la réserve, de prévoir des missions ponctuelles ou récurrentes, par exemple une difficulté liée à une tornade dans un lycée français qui mériterait une mobilisation de nos concitoyens auprès des enfants et des concitoyens : voilà le type même de mission qui pourrait être assumée par ces réservistes à l'étranger, Français et engagés.

Cet amendement a pour objet d'inscrire, au titre des activités permettant d'acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation, les activités de réserve. C'est une reconnaissance qui sera extrêmement utile pour ceux qui s'engagent pour la collectivité. En effet, au même titre que la réserve communale de sécurité civile, la réserve sanitaire ou militaire, les réservistes civiques, y compris ceux des réserves thématiques, doivent pouvoir bénéficier

rien ne justifiait que ces réservistes ne bénéficient pas du compte engagement citoyen, alors qu'il était ouvert à la réserve de la gendarmerie nationale : c'est une mesure de justice au regard de ceux qui s'engagent auprès de la police nationale. Enfin, en sens inverse, sont retirés les volontaires des armées, puisque ce sont des contractuels

commission a déjà adopté un amendement du Gouvernement visant à inscrire le volontariat de la réserve civile de la police nationale parmi les activités de volontariat permettant, dans le cadre du compte engagement citoyen, d'acquérir des heures

au motif qu'ils sont des contractuels et que leur activité ne peut être assimilée à un engagement bénévole. Monsieur le ministre, en réponse à l'une de mes questions, vos services m'ont confirmé que les contrats de volontaires ouvraient de plein droit l'accès au compte personnel de formation, sans passer par l'intermédiaire des heures de formation au titre du compte engagement citoyen- je ne doute pas que vous suiviez parfaitement,

Mme Christine Prunaud. L'engagement associatif représente souvent une forme d'élitisme social. C'est ce qui ressort des derniers rapports de France Bénévolat et d'études sociologiques. Si le secteur associatif s'en est rendu compte et tente d'attirer de nouveaux publics, il est tout aussi vrai que les dispositions prévues par l'article 8 vont dans le bon sens. Mais encore faudrait-il que ce congé soit rémunéré, et c'est ce que nous proposons par le biais de cet amendement. Le constat dressé par Le Mouvement associatif, fédération de 600 000 associations, révèle que, s'il n'y a pas à proprement parler de crise du bénévolat, la complexification des normes concernant les associations, associée à un caractère chronophage des postes de direction, conduit à des difficultés de renouvellement des responsables associatifs. De fait, occuper une responsabilité aujourd'hui dans une association nécessite du temps et, potentiellement, des ressources suffisantes pour pouvoir s'absenter occasionnellement du travail, ainsi qu'une formation solide pour mener à bien l'administration de la structure. En ce sens, l'instauration du congé associatif est une bonne chose, même si se pose la question de son applicabilité réelle.

À terme, c'est la question de leur renouvellement qui se posera. Or, si le bénévolat progresse, ses modalités ont évolué. Il est plus ponctuel, plus informel et se traduit moins par une implication collective durable, ce qui rend la conduite d'un projet associatif dans le temps plus difficile. Souvent, celui-ci repose sur un noyau dur de bénévoles très engagés, et les projets sont de plus en plus complexes. L'une des principales raisons de cette évolution réside dans le manque de disponibilité : le manque de temps est majoritairement invoqué par les personnes qui ne donnent pas de leur temps gratuitement. Si nous voulons réellement développer une culture de l'engagement à tous les âges de la vie, nous devons prendre en compte les évolutions du bénévolat et mettre en place un cadre favorable à l'engagement des actifs. C'est l'objectif visé par le congé des responsabilités associatives. Ce congé, qui est non pas une création, mais l'extension d'un congé existant et non rémunéré, est un moyen mis à la disposition des entreprises et des salariés pour mieux articuler les différents temps sociaux, concilier activité professionnelle et engagement bénévole au service de l'intérêt général. Le bénévolat et le soutien à l'engagement associatif profitent à tous. Les entreprises l'ont d'ailleurs bien compris et l'intègrent de plus en plus dans leur démarche de responsabilité sociétale, comme source d'« externalités positives », ne serait-ce qu'en termes de développement de compétences complémentaires de leurs salariés, d'ancrage territorial ou tout simplement d'image et communication. Ainsi, 60 % des grandes entreprises, 42 % des entreprises de taille intermédiaire, 36 % des PME et 20 % des TPE ont développé un partenariat avec une association. C'est pourquoi nous proposons le rétablissement de l'article 8.

y compris pour le lien national. C'est dans cette perspective que le Gouvernement souhaite que ce congé d'engagement, qui étend le dispositif du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, bénéficie à toutes les tranches d'âge, à tous les secteurs, à tous les actifs. Avec cette mesure, le Gouvernement ouvrait- je parle à ce stade au passé -un droit aux salariés, celui de consacrer du temps à leur engagement dans de bonnes conditions et dans un cadre sécurisé. Ce dispositif équilibré offre une possibilité nouvelle aux salariés sans pénaliser l'employeur.

de nouvelles inégalités entre les grandes et les petites entreprises : les petites entreprises sont pénalisées par les absences de leurs salariés et sont

fixer sur la participation aux organes d'administration et de direction d'une association, d'une part, et sur l'exercice bénévole des fonctions de direction et d'encadrement, d'autre part. Madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, faciliter l'engagement des responsables associatifs- c'est bien de cela qu'il s'agit de cela qu'il s'agit -, par ailleurs en activité professionnelle, est un réel enjeu pour notre société. Je rappelle que, pour 29 % des actifs non engagés, la conciliation d'une activité bénévole et d'une activité professionnelle est un frein.

C'est donc un besoin identifié depuis longtemps et depuis longtemps souhaité par nos partenaires associatifs. Permettez-moi de vous rappeler que le rapport sur l'engagement associatif des actifs, issu d'un groupe de travail conjoint entre le ministère de la ville l'association Le Rameau, qui m'a été remis en 2014, envisageait la création d'un congé rémunéré. Cette option n'a pas été retenue par le Gouvernement, même si certaines grandes entreprises, comme

La commission des lois a examiné sur le fondement de mon rapport, le 28 septembre dernier, le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

En revanche, la commission des lois a considéré que la réforme de l'appel à la générosité publique opérée par les articles 8 à 10 de l'ordonnance soulevait des difficultés. Cette réforme pose d'abord un problème de principe. En effet, alors que le Gouvernement n'était habilité par le Parlement qu'à modifier les règles relatives aux formalités imposées aux associations et fondations, il a modifié par cette ordonnance des règles qui s'appliquent indistinctement à des « organismes » quel que soit leur statut juridique. Or, en 1991, le législateur a volontairement retenu la notion d'organisme, ce qui regroupe les associations et fondations, mais aussi les mutuelles, les établissements publics, les fonds de dotation, voire de simples groupements de faits. Rappelons que, comme toute délégation de compétence, le champ de l'habilitation est d'interprétation stricte. Le fait que ces règles concernent essentiellement les associations et fondations n'est pas suffisant. En violation de l'article 38 de la Constitution, les modifications effectuées par ordonnance excédaient donc le champ de l'habilitation. légiférer par ordonnance sur ce sujet qu'il est particulièrement délicat à aborder. Si certaines modifications introduites par l'ordonnance sont bienvenues, comme je l'indique dans mon rapport, d'autres privent l'État de moyens de contrôle. termes de l'ordonnance, tous les organismes faisant appel public à la générosité ne sont plus tenus de déposer une déclaration préalable, ni même un compte d'emploi des ressources, pour justifier de l'affectation des ressources. Or la Cour des comptes et l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, qui sont habilitées à contrôler ces organismes, ont démontré dans leurs derniers rapports que certaines obligations élémentaires de publicité sont respectées par moins de la moitié des organismes soumis à cette législation.

Mes chers collègues, vous l'aurez compris, les deux amendements que j'ai déposés sur ces deux articles visent uniquement à traduire la position adoptée unanimement par la commission des lois la semaine dernière. Le

les pouvoirs qui sont les vôtres, le champ d'application de la loi concernant non seulement les associations et les fondations, mais aussi les organismes.

mesdames, messieurs les sénateurs, nombre d'associations aujourd'hui collectent les dons des particuliers toute l'année et sur leur site internet, ce qui n'était pas le cas, bien sûr, en 1991. Par ailleurs, les dispositions antérieures prévoyaient que ces campagnes d'appel à la générosité devaient nécessairement être menées à l'échelon national, ce qui, dans les faits, est loin d'être le cas, comme nous le constatons tous. L'ordonnance de simplification modernise donc ce cadre en faisant disparaître la référence à la notion de campagne et à sa portée nationale. La terminologie a été modifiée en conséquence. Ce qui compte désormais, c'est que l'appel à la générosité s'adresse bien au public, quelle que soit sa forme, privée ou publique, ou son caractère épisodique ou permanent. Votre amendement de suppression, madame la sénatrice, est motivé par le fait que les organismes concernés par ces dispositions ne seraient pas exclusivement des associations ou des fondations. que le Parlement a eu raison en 1991 d'établir une règle qui vaut quel que soit le statut de l'organisme concerné. Je ne puis donc pas être favorable à cet amendement, d'autant plus que, en réalité, les organismes faisant ces appels publics à la générosité sont aujourd'hui

à des aspects économiques. Enfin, tel qu'il est rédigé, l'amendement tend à créer entre ce type d'associations et les autres une discrimination quelque peu disproportionnée par rapport à l'objectif. En outre, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de ces obligations, ce qui affaiblit considérablement le dispositif. Les dispositions de votre amendement soulèvent une véritable question, qui n'a pas reçu à ce jour de réponse pertinente. Il serait donc extrêmement opportun que le Gouvernement se saisisse de ce sujet et propose au Parlement un dispositif

Nous en connaissons tous dans cet hémicycle. Par ailleurs, le dispositif proposé est totalement inopérant, car la caractérisation des associations susvisées ne s'adosse à aucune disposition législative ou réglementaire, comme vient de le dire Mme la rapporteur. Il faudrait donc les créer. Les préfectures seraient dans l'incapacité

cultuelles préfèrent utiliser le régime associatif de la loi de 1901. L'amendement tendait donc à imposer aux associations ayant un objet cultuel de se soumettre à la loi de 1905, alors que l'article 4 de la loi de 1907

lequel impose des sanctions en cas de non-respect des obligations imposées par la loi de 1905. Cela confirme ma conviction, et celle de la commission spéciale,

Ne vaudrait-il pas mieux rédiger une proposition de loi, que le Sénat examinerait avec attention, en se donnant le temps de l'analyse ? Cela me paraîtrait plus opportun

Il vise à soumettre les associations soumises au régime de la loi de 1901 qui entretiennent un lien direct ou indirect avec une autre association constituée pour l'exercice d'un culte aux dispositions de la loi de 1905.

L'option prise par le Gouvernement, notamment par le ministère de l'intérieur, que nous avons consulté, consiste davantage à faire oeuvre de pédagogie, en explicitant dans des guides réalisés avec l'appui des différents cultes, qui se sont associés,

a adoptée très largement en novembre 2014. Je rappelle qu'il s'agissait d'adapter le service civique aux besoins des sapeurs-pompiers. Près de deux ans après l'adoption par

Une telle possibilité nous permettrait de remédier à ce que l'on appelle la crise de l'engagement volontaire, ou crise de vocation. Beaucoup de chiffres circulent, mais tous vont dans le même sens : le nombre de sapeurs-pompiers volontaires ne cesse de diminuer. C'est l'ossature même de notre système de protection et de sécurité civile qui est menacée du fait de l'érosion des effectifs. Il faut impérativement inverser la tendance. Plusieurs initiatives ont d'ores et déjà été prises en ce sens. Les dispositions du présent article, tout comme notre proposition de loi, restée bloquée à l'Assemblée nationale, visent à effectuer un pas de plus dans cette l'une des difficultés que pose le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires est la longueur de la formation initiale, source de découragement et de renoncement. J'ajouterai que le volontariat doit davantage se féminiser et se diversifier, en intégrant les jeunes issus de la diversité. Cet article, tout comme ma proposition de loi, a pour objectif principal de répondre aux difficultés posées par la longueur de la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires et, en même temps, à la frustration des engagés de service civique, lesquels ne peuvent pas actuellement intervenir aux côtés des sapeurs-pompiers en opération. De plus, et dans tous les cas, ce service civique suscitera des vocations et pourra constituer un véritable levier d'engagement pérenne de jeunes en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Il s'agit de réamorcer la pompe du volontariat. La parole est à M. parole est à M. Joël Guerriau, sur l'article. L'article 9 est une excellente initiative, puisqu'il fait de l'engagement des jeunes, tant au sein des SDIS que de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, une réalité opérationnelle. L'engagement des sapeurs-pompiers volontaires est encadré par la loi de 2011. Les jeunes sapeurs-pompiers reçoivent une formation tout au long de l'année scolaire, durant quatre ans, généralement le mercredi ou le samedi, en fonction du rythme scolaire. Il existe aussi le dispositif des cadets, destiné aux collégiens et aux lycéens. Les jeunes sapeurs-pompiers volontaires forment un vivier de recrutement de 15 %.

très faible. Cela s'explique-t-il par la montée de l'individualisme et le recul des valeurs d'altruisme et d'entraide ou par un manque d'information des jeunes sur les possibilités d'engagement en matière de sécurité ? Depuis 2015, une convention conclue entre le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministère de l'intérieur permet à chaque élève de recevoir au cours de sa scolarité une formation aux premiers secours. Ces échanges permettent l'inscription de jeunes en tant que volontaires dans les services départementaux d'incendie et de secours et dans les centres de secours. Il faut admettre qu'il est rare que les jeunes de onze à dix-huit ans soient bien renseignés sur les possibilités qui leur sont offertes de s'engager dans la sécurité civile. Les missions accomplies par les sapeurs-pompiers paraissent souvent éloignées des centres d'intérêt des collégiens et des lycéens. et des lycéens. Ne serait-il pas plus intéressant de leur présenter davantage l'engagement volontaire et les modalités de la formation des jeunes sapeurs-pompiers, pour que cet article puisse être véritablement opérationnel ? Encore faudrait-il que l'information

En France, quelque 80 % des pompiers sont des volontaires. Nous constatons partout dans nos territoires une diminution significative du nombre des volontaires, lequel est passé de 207 000 en 2004 à un peu plus à 192 000 en 2013, soit une perte de 15 000 volontaires.

ne fonctionnait pas bien- il avait accueilli 400 volontaires entre 2010 et 2011, contre 150 en 2014 -, tout simplement parce que l'on ne laissait pas ces jeunes accomplir les fonctions qui correspondaient à leurs motivations. Ils n'avaient ainsi pas le droit d'aller en opération.